La séance est reprise en forme Sénac : la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est parvenu à l'adoption d'un texte commun. Ce qui n'est pas si fréquent. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits d'émission, gestion des finances publiques et des ressources humaines crédit non répartis action et transformation publiques le compte spécial Gestion du Patrimoine immobilier de l'État et la mission régimes sociaux et de retraite article qu'on s'spécial pension. La parole est à monsieur Claude nous, rapporteur spécial de la commission des finances pour les missions, gestion des finances publiques et des ressources humaines est parti, action et transformation publiques pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la mission sont des finances publiques et des ressources humaines et la principale mission du pôle économique et financier de l'État, l'année fiscale et la anis façon dédouane représentent les 3 quart de cet ensemble, le reste étant composé de diverses structures transversales ou d'État-Major. Les crédits de la mission sont stables en 2018 à environ 11 milliards d'euros d'une manière générale, les dépenses ont maîtrisé la programmation budgétaire et sincère et l'évaluation de la performance s'améliore après tout, ce sont les domaines où Bercy doit donner l'exemple. La masse salariale représente à elle seule 80 pourcent des crédits de la mission, c'est donc sur ce point que porteront l'essentiel de mes remarques. Cette année encore, ce sont les ministères économiques et financiers qui contribue le plus fortement à la réduction du nombre d'agents publics alors si pression 2450 emplois je rappelle par comparaison que les suppressions nettes sur l'ensemble du périmètre de l'État atteindront 1600 donc loi toutefois s'est efforcé atténuées depuis 2 ans. Auparavant, le schéma d'emplois était plus proche de 2000 emplois à temps plein par an. Cette inflexion à 2 raisons principales. Du côté de l'administration fiscale, comme l'année dernière 500 postes seront préservés, afin de préparer la mise en demeure du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, se rappelle qu'il s'agit d'une réforme très complexe, c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a choisi de la décalé à 2010. Du côté de l'administration des douanes l'exercice 2018 verra la création de 200 postes supplémentaires, faisant suite aux créations de 2007 et 2007, c'est d'abord la réponse à une série de crises ponctuelles, les attentats de 2015, puis le Brexit en effet 85 pourcent des liaisons routières entre le Royaume-Uni et le continent passe par la France.

le cycle de renouvellement des moyens maritime tous d'ailleurs à sa fin. Ceci dit, pour la nutrition fiscale comme pour la douane il y a pour ainsi dire de mouvements parallèles qui sont à l'oeuvre d'un côté les nouvelles priorités, donc je ne parlez et qui justifie les créations de postes, de l'autre, un chantier de plus longue haleine, celui de la rationalisation de leurs réseaux. Philippe compte plus de 4000 implantations et les regroupements se sont accélérées depuis 2 ans, 55 centres des impôts. Et 125 trésoreries rurales trop fragiles devrait fusionner l'année prochaine. Il en va de même pour les quelque 840 brigades et bureaux de douane. Service le peut pas fonctionner correctement. Avec moins de 4 ou 5 jours. Cependant si cette évolution est nécessaire, la concertation avec les acteurs locaux restent trop souvent défaillante, sa canne effraction a tendance à prendre des décisions seul, de son côté. De sorte que territoire peut à plusieurs services publics à la fois. Monsieur le Ministre, pourriez-vous donc prendre à cet égard, quelques engagements. Par exemple, est au minimum de ne pas arrêter, décision avant le vote des schémas départementaux d'amélioration et d'accessibilité des services au public prévue par la loi Meurtre d'ailleurs ou encore assurer une certaine prévisibilité lorsque les évolutions sont évidentes, par exemple, pour être alors et hospitalière ou l'adaptation à la nouvelle carte intercommunale. Maintenant, un mot rapide sur la mission crédit non répartis cette mission comprend de notation prévue par la LOLF afin de couvrir des dépenses qui ne peuvent être répartis au moment du vote de la loi qui lance ce montant atteint 100 même 4 millions d'euros, compte tenu de l'amendement du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale et la dotation de provisions relatives aux rémunérations publiques n'est plus le programme dépenses accidentelles. Et imprévisible et, quant à lui, majoré de 100 millions par rapport à 2017, le gouvernement justifie Monsieur le Ministre, cette majoration. Pas l'objectif de compenser partiellement la baisse du taux de mise en réserve des crédits par mission de 8 Si cette réduction de la mise en réserve, ça serait d'un plus grand respect de l'théorisation parlementaires des. Pourquoi, chers collègues. L'augmentation des crédits de cette mission qui échappent au principe de spécialité DD pense appelle toutefois cette remarque : nous serons vigilants, Monsieur le Ministre, quant à l'exécution des crédits non répartis au cours de l'année 2018 qui vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Thierry Carcenac, rapporteur spécial de la commission des finances. Pour sa minutes également. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, s'agissant de la mission gestion des finances publiques et des ressources du même je souhaiterais pour ma part, attirer l'attention du gouvernement sur 2 points particuliers : premièrement, l'organisation interne des services, la DGSI, on est prochaine plusieurs efforts majeurs auront un impact systémique sur le travail des agents le prélèvement à la source, la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des foyers, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique de l'impôt sur la fortune immobilière ou encore la suppression en 2019 du CIC à ce stade, nous constatons peu d'anticipation et un certain attentisme sur les conséquences de ses décisions, mais peut-être pourriez-vous nous rassurer sur les orientations prévues Monsieur le Ministre, deuxièmement les grands chantiers informatiques qui en est l'objet d'investissements importants. Les ministères économiques et financiers représentent 15 pourcent des projets informatiques de l'État et 20 pourcent des dépenses, il faut le souligner ceci n'accuse pas ou plus le surcoût retard excessif par rapport aux autres ministères, ceci dit, c'est avant tout parce que les projets les plus importants sont terminées, donc ils ont échoué, je vous rappelle à cet égard le précédent de l'opéra de l'opérateur national de paix menés en pure perte, avant d'être interrompu en 2014 plusieurs projets actuels, notamment en matière de gestion de ressources humaines vise seulement à réparer les conséquences de cet accident pour réussir les grands projets informatiques de demain, les pistes sont claires : une gouvernance renforcée au niveau interministériel, une meilleure mutualisation des projets, une réduction de la dépendance aux prestataires extérieurs et Coralie hâtivement une meilleure expertise en temps. Monsieur le Ministre, quelles sont les conséquences du décret du 21 novembre 2017 relatifs à la Direction interministérielle de la transformation publique et à la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. L'un des grands enjeux pour l'avenir concerne d'ailleurs la capacité de recruter et de fidéliser des profils de haut niveau dans les métiers du numérique, je présenterai 2 ans demande permettant d'aborder cette question essentielle pour l'État et les administrations de réseaux de la mission. On passe maintenant au compte d'affectation spéciale Gestion du Patrimoine immobilier de l'État ne représente que 10 pourcent de la dépense immobilière de l'État, le reste étant par différentes missions du budget général, soit 44 programme il incarne pourtant l'État propriétaire est constitué de vecteur budgétaire de la direction de l'immobilier de l'État, il participent du principe essentiel de 10 fonctions entre l'État propriétaire et les ministères occupants je ferai demain, remarque d'abord en constat : l'intégration des dépenses d'entretien lourd de l'ancien programme 309 a pu se traduire par une modification de dépenses du compte, la part des dépenses de fonctionnement, a certes progressé au détriment des peu dépenses d'investissement, mais celle-ci diminue de 30 pourcent en 2018 par rapport à 2017 j'aimerais, monsieur le ministre, connaître votre analyse sur cette évolution ensuite un décryptage la instabilité des crédits du compte par rapport à 2017 est en trompe-l oeil en raison d'une opération exceptionnelle prévue en 2018, les établissements d'enseignement supérieur d'aménagement sur le plateau de Saclay feront exception à la mutualisation des produits de cession décidée lors des précédentes lois de finance l'intégralité sera donc reversée au ministère de l'enseignement supérieur ainsi neutraliser les crédits immobiliers effectivement disponibles sur le compte, diminue de 12 pourcent par rapport à 2010, ce recul contraste avec les nouvelles orientations dans la pop dans la politique immobilière a besoin avec notre ancien collègue sénateur Michel Bouvard nous avons proposé une feuille de route pour renouveler la gestion de l'immobilier de l'État, 10 ans après la création du compte, il nous faut te évoluer de la retenue de la rationalisation initiale à la recherche d'une meilleure valorisation du Patrimoine immobilier, pas forcément par des cessions d'ailleurs il me semble que plusieurs éléments semblent annoncer une nouvelle orientation après la création de la direction immobilière de l'État, c'est pourquoi monsieur le ministre, j'aimerais connaître vos projets en la matière, je terminerai mon propos en évoquant le grand plan d'investissement, la participation au du compte d'affectation spéciale est artificielle, dès lors qu'il s'agit de crédits qui étaient déjà prévus désormais précédente telle n'est pas le cas de la nouvelle mission du budget général action et transformation publiques l'intégralité de ses crédits doit participer au grand plan d'investissement au titre de la rénovation des cités immobilière et du Fonds pour la transformation de l'action publique, un montant de 1 milliard 7 d'euros est prévu pour les 5 prochaines années, cependant la démarche demeure à ce stade, essentiellement programmatique, puisque l'essentiel des crédits devraient être ouverts à compter de 2020, surtout en vertu du principe de réallocation décret du grand plan d'investissement des crédits prévus dans la programmation plus Rennes il faut conclure, pourront être réallouer entre les différentes actions prend le président de la commission des finances vous propose l'adoption des crédits de la mission, en précisant que nous resterons vigilants sur les évolutions à venir, à titre personnel, compte tenu des modifications adoptées par la majorité sénatoriale de la commission, je ne pourrais les adopter. Merci, Merci, la parole est à Madame Sylvie Vermeillet, rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes également. Monsieur le président Monsieur 2 ministres Madame messieurs les rapporteurs mais, chers collègues, je relève le défi de vous présenter un rapport de 65 milliards d'euros en 5 minutes, avaient constitué des régimes spéciaux de retraite 6,3 milliards versés par l'État pour équilibrer certains régimes spéciaux SNCF, RATP marins mines etc et puis les pensions civiles et militaires 58,4 milliards d'euros au compte d'insectes à Sion spéciale pension concernant les régimes spéciaux, le nombre de cotisants étant très inférieur au nombre de retraités, la contribution de l'État pour en assurer l'équilibre a fortement augmenté entre 2006 et 2012, puis baissé entre 2015 et 2017 en 2018 la contribution augmente de 0,4 pourcent sous l'effet en année pleine de la revalorisation des pensions, début octobre, le ratio démographique de la SNCF et de la RATP se dégrade encore, et le déficit sera supérieure aux économies des régimes fermé mais sans tenir compte d'un éventuel retour de croissance la subvention d'équilibre de l'État représentent 68 pourcent du financement des retraites des régimes spéciaux, pour mémoire, l'ensemble des régimes spéciaux, compte 500000 actifs pour 1 1000000 100 1000 pensionnés et le régime général compte 18 millions d'actifs pour 15 millions de pensionnés, les régimes spéciaux ne se singularise pas seulement par le déséquilibre démographique des différences institutionnelles et économiques persistent, comme l'âge de départ en retraite de 50 puis 52 ans, pour le personnel roulant de la SNCF, la RATP et 55 8 57 ans, pour les autres, contre 62 ans d'âge légal en dehors de toute réforme le déséquilibre des régimes spéciaux, ce serait quand même réduits pour la SNCF, il serait passé de 4 à 2,5 milliards annuels d'ici 2050 les réformes successives de ces dernières années, la tenue, mais le déficit perdure et l'appel à la solidarité nationale est toujours nécessaire, c'est une des questions de la prochaine réforme celle de financement mais aussi celle de l'équité et c'est une question économique, enfin, puisque beaucoup dépendra de la capacité de la SNCF, a relevé le défi de l'ouverture à la concurrence concernant le compte d'affectation spéciale pension 58,4 milliards d'euros, pour les pensions civiles et militaires de la fonction publique d'État 3,3 pourcent pour les ouvriers établissements industriels de l'État 3,2 pourcent pour les pensions militaires d'invalidité, victimes de guerre et du terrorisme, les dépenses en très forte hausse depuis 25 ans sont passé de 19,1 milliards en 90 à 58,4 milliards en 2018 le nombre de bénéficiaires a doublé le niveau des pensions des entrants et globalement supérieurs aux pensions en cours, mais le taux de remplacement tend à baisser sous l'effet des réformes successives pour 2018, le gouvernement ne revalorisera pas les pensions pour une économie d'environ 137 millions encadre prise de l'inflation, l'économie sera encore supérieur, les pensions brutes vont perdre en pouvoir d'achat, les pensions être plus en quart car la CSG va augmenter un milliard pour les seuls fonctionnaires de l'État, du côté des recettes le gel indiciaire et le report du PPCR décidée par l'État vont soulager la masse salariale mais se traduiront par moins de recettes pour le compte d'affectation spéciale de de 243 millions d'euros de recettes qui ne sont pas de budgéter. Le solde excédentaire du compte d'affectation spéciale atteindrait 7,6 milliards fin 2018 très supérieur aux besoins de trésorerie, rappelons que la Cour des comptes, le trouver excessif dès 1,6 milliard, le ministère des Finances a abandonné d'expliquer qu'il s'agit de financer les déficits prévisionnels à court terme puisque le solde cumulé devrait atteindre plus de 25 milliards vers 2030 hors bilan les engagements financiers de l'État au titre des retraites ont été brusque le relevé dans le compte général de l'État, passant de 1535 milliards fin 2015 à 2139 milliards actuellement en raison du changement de modèle de prévision et du taux d'actualisation qui devient négatif, je m'interroge sur la cohérence avec le scénario de retour à la croissance en conclusion quelques interrogations : faut-il continuer de sur-financier le casse en abaissant le niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population et validé une baisse très significative des taux de remplacement. Deuxièmement, réformer les retraites suppose de réformer la politique des ressources humaines de l'État cet état très employeur doit devenir mieux employeur si l'on veut que travailler plus longtemps et du sens enfin puisque le processus de réforme est en cours, il faut souhaiter que le Parlement soit pleinement informé des avancées des travaux de Jean-Paul Delevoye Haut-commissaire à la réforme des retraites, l'idée d'une égalisation des rendements je conclus les cotisations et populaire, mais je rappelle que globalement cette égalisation a beaucoup progressé, si l'on compare les différentes générations les écarts qui demeurent sont principalement liées à des conditions de travail inégal ou à des conditions de vie différente, comme pour les gendarmes, les militaires, en général, il sera compliqué de vouloir un rendement de cotisation égale pour un effort inégal. Merci, cher collègue, je pense qu'il faut s'arrêter parce que sinon on déborde. La commission des finances vous propose d'adopter les crédits de la mer régimes sociaux et de retraite, éducation. Merci, la parole est à René-Paul Savary, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur spécial, chers collègues, je veux intervenir c'est tombé en complément de ma collègue Madame Vermeillet au de la commission des affaires sociales, en appuyant mot discours effectivement sur des propositions qui, sur moins de chiffre, c'est normal, commission des affaires, les finances d'un côté, commission des affaires sociales de l'autre, simplement effectivement nos missions sur le le compte d'affectation spéciale ou sur la mission particulière régimes sociaux de retraite porte sur 68 milliards c'est un petit bout de la partie des retraites obligatoires qui porte sur plus de 138 milliards, sachant que l'ensemble des retraites a été complémentaires, c'est plus de 310 milliards donc sont quand même des sommes significatives et donc le montant de 68 milliards ne couvrent d'ailleurs ni l'ensemble des dépenses du régime de retraite de la fonction publique, ni même l'ensemble des autres régimes spéciaux et des masses financières importantes, comme la Cnracl pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ou même le régime des industries électriques ou gazières ne sont pas concernés par ces missions budgétaires alors que la réforme annoncée promet qu'à terme, un Euro cotisé devra rapporter la même chose, quel que soit le statut du cotisant ou le régime dans lequel il a été versé ces régimes spéciaux soulève 3 questions premières quel avenir, quel avenir pour les règles de départ à la retraite qui demeurent éloignées du droit commun, si elle semble indissociable de la carrière de militaires, par exemple, elles apparaissent toujours contestable pour les assurés des régimes de la SNCF et de la RATP par exemple le de même 2ème question de quel avenir pour le mécanisme de contribution employeur au sein des régimes de la fonction publique qui ne permet pas actuellement de distinguer la part patronale de l'employeur public d'une part, la compensation en déséquilibre démographique de ces régimes, d'autres pas, et enfin le financement de dispositifs de retraite dérogatoire si un Euro cotisé Édouard rapporté la même chose, il ne peut substituer de différences dans le niveau de la participation employeur, ce qui implique d'avoir des taux de rendement similaire entre tous les régimes de retraite et ce point sera déterminant pour la réforme de la retraite à venir enfin quel avenir pour le paysage aussi morcelé, des retraités, ses quelques 35 régimes de base, alors que le coût de gestion des 310 milliards d'euros de prestations. Retraites de base et complémentaires célèbre entre 5 et si il y a. ça doit nous interpeller, c'est le défi qui nous attend en 2018 avec cette réforme, comprendre la complexité du système de retraite pour mieux le réinterroger en profondeur, quel dispositif de solidarité : souhaitons-nous conserver comment les valoriser en terme de points ou d'Euro, alimentant les futurs comptes notionnels, en attendant le lancement de cette réflexion à laquelle le Sénat participera pleinement notre commission a émis comme la commission des finances, un avis favorable à l'Inde option des crédits de ces 2 missions budgétaires, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Pour 3 minutes. Monsieur le président, monsieur Ministre, chers collègues, avant de présenter rapidement leur programme 148 j'ouvre une parenthèse sur la gestion de la masse salariale de l'État, le président de la République a annoncé sa volonté de supprimer 120000 équivalents temps plein durant son quinquennat dont 50000 dans la fonction publique d'État 70000 dans la fonction publique territoriale, or ce PLF prévoit une suppression nette 2600 équivalents temps plein dans la fonction publique de l'État, dont seulement 324 dans les ministères, ce qui est très insuffisant pour respecter cet engagement, nous pouvons donc légitimement nous interroger sur la méthode envisagée par le gouvernement pour respecter les objectifs fixés en ce qui concerne la fonction publique territoriale de l'État n'a pas à vocation à dicter le schéma d'emplois des collectivités territoriales, cependant, force est de constater qu'une réduction des dotations de l'État aux collectivités les oblige à réorganiser leurs services, voire à diminuer les services au public, il sera intéressant de suivre les travaux du comité action publique 22 chargée d'examiner les pistes d'évolution du service public et de ses effectifs concernant programme 148 Fonction publique mais il ne concerne que la fonction publique de l'État et comprend 3 actions interministérielles qui complètent les initiatives ministérielles, la formation, l'action sociale et le développement de l'apprentissage, il est doté de 239,11 millions d'euros, soit une baisse de 0 43 pourcent par rapport à 2017

la subvention Aléna, baisse de 2,75 pourcent par rapport à 2017, en revanche, la subvention 5 ira progresse de plus de 10 pourcent pour poursuivre les efforts entamés à la rentrée 2017 et satisfaire les besoins de recrutement d'attaché d'administration des ministères plus 98 élèves accueillis à la rentrée 2017 de plus un effort significatif est consenti pour les actions spécifiques de formation interministérielle plus 24 pourcent par rapport à 2017 les plateformes régionales d'appeler interministériel à la gestion des ressources humaines, situées dans les préfectures de région joue un rôle essentiel pour développer et coordonner ces actions de formation, j'avais l'an passé, préconiser le renforcement de leur visibilité et la clarification de leur mission et gouvernance

les crédits consacrés au développement de l'apprentissage, baisse de près de 3 millions d'euros, ce qui est en contradiction avec l'objectif d'atteindre le seuil de 10000 apprentis recrutés dans la fonction publique d'État, le Fonds Innovation RH, créée en 2017 et pérenniser à hauteur de 1 1000000 d'euros afin de soutenir les initiatives innovantes des ministères

et le fonds des systèmes d'information RH à hauteur de 1,83 millions pour ouvrir aux agents publics, le portail informatique du compte personnel d'activité concernant ce dispositif et notamment le compte personnel de formation il clarifie la formation et permet aux agents de construire un parcours professionnel cohérent cependant sa réussite dépendra de la manière dont les agents publics se l'approprier en or, on constate qu'ils ont des difficultés à actionner leur droit à la formation, les employeurs publics sont appelés à jouer un rôle majeur dans sa mise en oeuvre, cependant il manque d'informations sur ce fonctionnement et monsieur le ministre, il me semble urgent d'organiser, de coordonner les actions de sensibilisation au plus près des employeurs et des agents publics sans cet effort de pédagogie, le compte personnel d'activité pourraient connaître les mêmes difficultés que le droit un visuel à la formation, je conclus en disant que la commission des lois a adopté les crédits du programme 148 je vous remercie. Chers collègues, donc nous passons à l'expression des groupes qui vaut, explications de vote, je le rappelle, donc, la parole est Hamas dames Josiane Costes du groupe RDSE pour 6 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, l'émission que nous examinons à présent porte sur la politique de l'État employeur, par le biais de la mission en gestion des finances publiques et des ressources humaines et de la mission concernant les régimes sociaux et de retraite, ainsi que sur la et de retraite, ainsi que sur la politique de l'État propriétaire par le biais du compte d'affectation spéciale Patrimoine immobilier de l'État, avec près de 2 millions de fonctionnaires, l'État étonnant ployant de 1er plan et la gestion de son personnel, a une importance cruciale, avec des implications pour l'efficacité de l'administration, la qualité des services publics, le développement économique si le gouvernement prévoit une réduction des effectifs en 2018 elle demeurera tout de même limité en dessous de 2000 suppressions de postes, les grandes masses d'effectifs par ministère resteront stables avec les 3 quarts de la fonction publique d'État, répartis dans l'éducation nationale, l'intérieur et les armées des ministères connaîtront toutefois de fortes baisses d'effectifs, comme le travail, la santé et le logement, l'analyse de la mission régimes sociaux et de retraite et du combat affectations spéciales relatif aux pensions des fonctionnaires appellent les commentaires suivants si les retraites des régimes spéciaux restent encore subventionnés dans des proportions importantes, le besoin de subventionnement tend à décroître et là, la situation de ces régimes au demeurant très diversifiée tant à converger avec le régime général, de leur côté le solde du C. A. S. pensions des fonctionnaires est nettement excédentaire, même si cet excédent se réduit en 2018 sa situation paraît satisfaisante au regard de celles du régime général, en revanche, le rapport spécial n'étant en lumière des insuffisances et des points à améliorer dans la gestion des ressources humaines de l'État, ainsi les déploiements de programmes informatiques crée souvent des difficultés importantes, les difficultés rencontrées dans leur mise en place, comme par exemple l'échec du logiciel de paie désormais Louvois entraîne des retards et des surcoûts parfois importants, il apparaît donc essentiel d'améliorer la situation des administrations dans ce domaine, cela passe aussi par des organisations repenser une meilleure gestion des ressources humaines et des carrières à une meilleure utilisation des compétences au sein des services et une meilleure négociation des contrats de fournitures et de services avec les prestataires extérieurs, donc de la fonction achat de l'État, d'autres risques ont été soulignés qui sont liés à l'qui sont liés à la mise en oeuvre par la direction générale des finances publiques des réformes prévues dans ce projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative, que nous examinerons prochainement nouvel impôt sur la fortune immobilière en remplacement d'une Yacef prélèvement à taux unique sur les revenus d'épargne révision des bases locatives et surtout mise en place du prélèvement à la source, le pilotage de ces réformes lorsqu'elles auront été votée sera déterminant dans le succès de leur mise en oeuvre, j'en viens maintenant à la politique de l'État propriétaire les informations budgétaires relatives aux pratiques Patrimoine de l'État sont retracés dans le C. CCAS PIE et sa gestion est confiée à la direction de l'immobilier de l'État, rattaché à la DG les principales évolutions de 2018 selon la contribution du compte spécial au grand plan d'investissement décidé par le 1er Ministre des recettes liées à la cession du Patrimoine immobilier des établissements d'enseignement sur supérieur et de recherche qui quittent leurs anciennes simple implantation pour rejoindre le plateau de Saclay, au-delà de ces nouveautés, le principal enjeu de la gestion du Patrimoine de l'État et la définition d'une stratégie patrimoniale à long terme, l'État doit répondre à un double impératif préserver et valoriser un Patrimoine historique de grande valeur qui représentent une richesse incomparable pour la nation, rénover et développer le Patrimoine pour un usage optimal pour les administration occupante ainsi la rénovation des cités administratives sur l'ensemble du territoire est une priorité des bâtiments de qualité fonctionnelles écologique auront également un impact positif sur le travail des administrations c'est l'objet de la mission action et transformation publiques que nous examinons conjointement avec l'émission compte cette cette émission porte en particulier sur la rénovation des bâtiments administratifs, le programme 348 finance ainsi la rénovation des sites occupés par plusieurs services de l'État ou de ces opérateurs, la mission comporte également le font pour la transformation de l'action publique au programme 349 chargé de financer le coût supplémentaire initial de l'engagement des réformes, le gouvernement a fort affirmé sa volonté de moderniser le fonctionnement de l'administration avec le projet action publique 2022, qui n'est pas sans rappeler les projets des gouvernements précédents RGPP MAP, la réforme de l'État et probablement aussi ancienne que l'État lui-même, toutefois j'accueille favorablement cette initiative, à condition qu'elle associe pleinement les fonctionnaires et l'ensemble des acteurs publics, enfin les crédits non répartis concerne les dépenses accidentelles et imprévisibles, tels que la compensation partielle de la hausse de la CSG dans la fonction publique à hauteur de 3 milliards d'euros, ce geste en faveur des fonctionnaires dans le pouvoir d'achat stagne depuis plusieurs années à Paris, bienvenue en conclusion sur ces 4 missions et ces 2 comptes Pessiot dans les heures, dans les enjeux, ils sont importants reste assez technique et difficile, a détaillé en quelques minutes de discussion, ainsi que sur l'article 55 terre rattaché à la mission, le vote des membres du groupe RDA ce sera globalement favorable. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Didier Rambaud la République en marche pour 6 minutes. monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons-les les crédits de missions qui ne sont pas les moins passionné, à commencer par la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines, qui comprend notamment le budget Fonction publique je souhaite m'arrêter sur ce budget moins pour commenter les chiffres, les rapporteurs, l'ont déjà fait et bien fait, mais pour insister sur les orientations du gouvernement en la matière, qui me semble aller dans la bonne direction, bien sûr, le groupe la République en marche soutient pleinement un gouvernement qui a fait de la sincérité budgétaire, un de ces aiguillon dès l'été dernier, la Cour des comptes a mis en évidence que le plan de revalorisation des carrières des fonctionnaires n'étaient pas financés dès lors que faire, laisser filer les déficits publics et je ne reviens pas sur les enjeux politiques d'un passage durable sous le seuil de 3 pourcent ou en reporter l'application, je ne dis pas que la gestion des carrières des agents de la fonction publique est négligeable mais je conteste l'attitude de faire des promesses non financées à celles et ceux qui font vivre nos services publics, les perspectives de carrière, décidément, n'ont jamais fait bomber nagent avec les impasses budgétaires. J'ai aussi, bien entendu, notamment en commission des finances, les griefs que certains adressée au gouvernement sur le rythme jugé trop timide de réduction des effectifs, mais je m'étonne de ne pas avoir entendu des propositions précises à ce sujet, notamment en matière de fonction publique territoriale, nous saluons-les mesure courageuse prise par les ministres, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, à savoir le gel du point d'indice et l'instauration à l'article 48 du PLF pour 2018 dans les jour de carence pour les agents publics sur le point d'indice au-delà du gel, il pose la question de la centralisation sans doute excessive de la rémunération des fonctionnaires, mais aussi de la prise en compte du mérite sur le jour de carence, le dispositif a été mis en place entre 2012 et 2014, il s'agit d'une mesure d'égalité avec les salariés du secteur public, privé, mais aussi un dispositif de lutte contre l'absentéisme qui peut, qui peut nuire à la qualité du service public et qui n'est pas neutre pour les finances publiques, j'assume de dire qu'un certain nombre de dispositifs dérogatoires et je ne parle pas du statut ne sont plus adaptés et doivent être sinon réformer au moins évalué, à commencer par notre haute fonction publique, l'action publique ne se transforme pas par saccades, le gouvernement a donc décidé d'innover à travers le comité action publique 2022 au mois d'octobre avec une triple exigence qualité du service public pour les usagers, amélioration des conditions de travail des agents publics, maîtrise des dépenses publiques et donc des prélèvements des prélèvements obligatoires pour les contribuables en tant que parlementaires, nous avons un rôle à jouer comme partie prenante que comme passeur pour faire connaître cette initiative dans nos territoires jusqu'au mois de mars 2018, c'est le temps du diagnostic à partir d'avril, ce sera le temps de la mise en oeuvre opérationnelle, j'insiste sur la méthode originale, notamment à travers le forum de l'action publique qui implique agent public et usagers et qui permettra de faire remonter les préoccupations et les propositions du terrain, on ne réforme plus l'État, comme en 1967 ou 1997, car les Français ont changé et ont des aspirations légitimes de participation et d'évaluation de leurs services publics, par Internet, s'agissant d'Internet, je salue le volet transformation numérique de l'administration qui traduit les engagements du président de la République, l'objectif d'avoir 100 pourcent des démarches administratives dématérialisées d'ici 2020, 2 le développement d'un État plateforme développant de nouveaux services numériques de qualité, la conduite d'une utilisation optimale des données publiques sont d'excellente nouvelle la dématérialisation n'est pas un recul du service public, au contraire, elle traduit un engagement au plus haut au niveau de l'État de faire en sorte que l'égalité des Français devant le service public soit une réalité plus d'efficacité et moins de dépenses publiques et moins de stress et de migraine pour les Français, ces mesures devraient je crois nous rassembler sur l'ensemble des banques, des banques, je vais pas détailler plus avant le programme ambitieux du gouvernement, ce qui sera sans nul doute fait par le ministre, le Sénat peut pleinement vous accompagner dans cette démarche de transformation à travers des missions d'information de consultation locale des rencontres avec les usagers, les élus et les agents cette maison que je suis en train découvrir est en pointe sur les innovations technologiques et techniques et cette expertise pourrait être un appui précieux pour le gouvernement. Le groupe, la République en marche se prononcera donc favorablement à l'adoption des crédits d'émissions en discussion commune. Merci, cher collègue, la parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, contrairement aux années précédentes, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une discussion commune de la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines et de la mission régimes sociaux et de retraite, ce qui n'est pas obligatoirement des plus judicieux, concernant l'évolution pour 2018, des crédits de la mission régimes sociaux et de retraite, la réduction des crédits des régimes spéciaux suit celle de l'avait baisse du nombre des cotisants, la contribution de l'État au rééquilibrage des comptes spéciaux est en légère diminution également, enfin les négociations des conventions d'objectifs et de gestion 2018, 2021 poursuivent la réduction de 15 pourcent des dépenses de fonctionnement et de 2 5 pourcent des effectifs par an au détriment de la qualité des conditions de travail des personnels, ce que nous condamnons, alors que la refonte des régimes spéciaux de retraite était annoncée pour 2018, il semblerait que le gouvernement et reculer son projet en attendant la future et forme des retraites annoncée pour 2018 et finalement décalé en 2019, toujours est-il que la pension moyenne des fonctionnaires civils et des militaires a diminué à cela s'ajoute la décision du gouvernement de décaler la date de revalorisation des pensions, créant ainsi une année blanche pour les fonctionnaires en matière de revalorisation pour 2018 et aggravant, par conséquent, la baisse de leur pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat encore rêver par la hausse de la CSG de 1,7 points dont les mesures de compensation annoncées par le ministre sont toujours aussi opaque concernant les fonctionnaires, les crédits de la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines s'inscrivent dans cette logique, 10 ans après la mise en place de la révision générale des politiques publiques, le gouvernement poursuit les coupes budgétaires élu suppressions massives de postes, alors que les Paradise Papers ont révélé l'importance de renforcer les moyens de l'administration fiscale et douanière pour lutter contre la fraude et contrôler l'optimisation fiscale, le gouvernement maintient les services en situation de sous-effectif chronique, vous avez assuré, Monsieur le Ministre, qu'il est possible, je vous cite, de transformer le pays et d'assurer un meilleur service public avec moins d'argent, mais avec des services informatiques et numérique plus performant, mais n'oublions pas que la fermeture des guichets physiques pour motif d'économie laisse encore beaucoup de personnes au bord de la route et peuvent donc être un nouveau facteur d'exclusion sociale, le défenseur des droits, dans son rapport sur l'accès au droit, a mis en exergue quelques statistiques établissant un lien entre non-maîtrise du numérique et les difficultés d'accès au public, la vigilance s'impose enfin je conclurai par le vote de l'Assemblée nationale devait de l'amendement rétablissant la journée de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires non seulement une note publiée le 10 novembre par l'INSEE a démontré que l'existence de ce dispositif dans la fonction publique entre 2012 et 2014 n'a pas significativement modifié la proportion d'agents de la fonction publique de l'État absent pour raisons de santé, mais encore cette mesure fait avéré contre-productive en effet si les absences pour raisons de santé, de 2 jours ont diminué les absences d'une semaine à 3 mois ont augmenté durant cette période, le rétablissement du jour de carence a été justifiée par mesure d'équité entre secteur privé et secteur public mais les 2 tiers des employées du secteur privé, privé, bénéficiaient d'une couverture totale de jour de carence en 2009, en conclusion, le gouvernement s'attaque à notre modèle de fonction publique à la logique même de service public mais cher collègue en réduisant ses moyens ceux : effectifs et en rapprochant les règles de celles du privé, pour toutes ces raisons, nous voterons contre les crédits de ces 2 missions, je mer. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Claude Malhuret pour le groupe, les indépendants pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 missions examiner ce soir, gestion des finances publiques et des ressources humaines, action et transformation publiques et régimes sociaux et de retraite. Les évolutions liées à la première mission nous semblent aller dans le bon sens, des effectifs des ministères économiques et financiers est réel et doit être salué cet effort doit être un exemple pour les autres ministères et pour la sphère publique dans son ensemble, un service public diligents et de qualité est possible, avec moins de fonctionnaires, c'est l'occasion de saluer ici le sens du service de notre fonction publique, c'est son honneur que d'avoir traversé les réformes successives de la RGPP à la MAP en adaptant son action pour servir avec la même efficacité et le même dévouement des effectifs réduits n'enlève rien à cette excellence, bien au contraire. Le groupe, les indépendants soutient donc le président de la République dans sa démarche de suppression de 120000 postes de fonctionnaires sur la durée du quinquennat. Nous espérons néanmoins que la trajectoire de maîtrise des effectifs sera alignée avec cet engagement, les prévisions de l'année 2018 semble d'ores et déjà trop timide pour espérer atteindre les objectifs de masse salariale fixée par le gouvernement. Ces diminutions de postes de fonctionnaires doit s'accompagner d'une réflexion d'ampleur sur les secteurs de l'action publique que nous attendons sanctuarisés ou en force comme la sécurité, la défense ou la justice, sur une réflexion également sur les dépenses in efficiente ou peu utiles sur la nature de l'État que nous voulons c'est missions essentielles son périmètre, ses modes d'action. Nous espérons que la nouvelle mission c'est la deuxième examiner ce soir la mission action et transformation publiques obtiendra des résultats à la hauteur de son intitulé volontariste, il serait extrêmement décevant qu'elle se limite à soutenir une revue de dépenses telles que celle que nous connaissons depuis quelques années à l'effet l'efficacité plus que discutable. Le comité action publique 2022 que vous pilotez demain devrait être ambitieux dans son approche de la révision des politiques publiques, il devra surtout s'affranchir d'un certain nombre de tabous qui ont vidé de leur substance les initiatives des précédents gouvernements. Par exemple, il ne pourra pas faire l'économie d'une réforme d'envergure de la fonction publique et du statut des fonctionnaires ainsi que de la simplification des normes et des procédures dans le domaine de la mobilité des instances de représentation de la grille salariale et des retraites des fonctionnaires, la Cour des comptes, rappelle d'ailleurs régulièrement leur nécessaire rapprochement avec le régime du secteur privé. Les retraits sont justement l'objet des crédits de la 3ème, mission que nous examinons aujourd'hui ceux de la mission régimes sociaux et de retraite correspond aux subventions d'équilibre que l'État verse à divers régimes spéciaux de retraite. Dans l'autofinancement et rendues impossibles par un déséquilibre démographique de plus en plus insoutenable. Ces subventions s'élève ta 6,3 milliards d'euros dans le PLF 2018, principalement entre les régimes des transports terrestres des marins et des mineurs. Nous devrons réfléchir à une réforme profonde à une refonte profonde de ces régimes spéciaux de retraite dont l'équilibre financier est rompu depuis l'origine, et dont le modèle n'est pas tenable sur le long terme. Le président de la République et le 1er ministre se sont engagés à mener à bien cette réforme d'ampleur des régimes de retraites, avec l'instauration d'un système universel, nous soutiendrons ces efforts vers la mise en place d'un système plus équitable, plus juste et plus solides financièrement. Pour conclure, le groupe des Indépendants républiques et territoires soutiendra le gouvernement dans sa volonté d'améliorer les services publics, de renforcer notre fonction publique et de moderniser l'action de l'État au service de nos concitoyens, nous voterons donc les crédits de ses missions avec un regard particulièrement vigilants sur les résultats concrets du processus action publique 2022, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de commission, mesdames et messieurs les rapporteurs mais chers collègues aborder un budget de cette ampleur dans un temps à peine supérieur à 2 chansons de feu Johnny Hallyday relève du du en effet, nous débattons aujourd'hui de mission qui font et feront l'objet de chantier de transformation important: la gestion des finances publiques et des ressources humaines, ainsi que les régimes sociaux et de retraite, la 1ère de ces missions, comprend l'essentiel des moyens de fonctionnement et d'investissement des ministères économiques et financiers qui apparaissent stables par rapport à 2017, ce qui est à souligner : nous saluons l'effort du gouvernement d'assumer une réduction des effectifs, tout en accompagnant la modernisation des équipements, la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et des droits indirects qui sont les 2 principales directions concernées assument leur mission avec 1450 effectifs en moins, cet effort est particulièrement important pour cette dernière, confronté à de nouvelles missions, suite au rétablissement des contrôles induit par la menace terroriste, elle concourt à l'objectif de maîtrise de l'emploi public, grâce au redéploiement des moyens humains et à la transformation numérique, nous saluons également la rupture avec la logique précédente durable, le gouvernement engage une réflexion qui nous paraît plus pertinente en interrogeant en profondeur l'ensemble du périmètre de l'action publique, l'État doit se poser les bonnes questions : quelles missions doivent aujourd'hui exercé la puissance publique, comment, avec quels moyens il existe un panel de solutions et le gouvernement a d'ores et déjà fait preuve d'un certain courage en réintroduisant, nous pensons que ça la différence de nos collègues, le jour de carence pour les personnels du secteur public, notre groupe de défend depuis des années, cette réforme, qui doit être considérée comme un gage d'équité entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public, quelques questions demeurent aujourd'hui quelle sera la trajectoire de diminution du nombre d'agents de la fonction publique. Pour nous, la maîtrise de la masse salariale publique exige une réforme d'envergure de la fonction publique, en parallèle, les crédits d'investissement visant à conduire les projets informatiques et numériques nécessaires à la modernisation de l'administration sont en hausse de 52 millions d'euros et ce sont 700 millions d'euros, dont 200 millions dès 2018 que vous consacrez à la transformation numérique de service public. Je me permettrai tout de même une mise en garde que cette dématérialisation ne ou n'accentue pas la fracture territoriale, n'oublions pas les administrés les plus vulnérables qui vivent parfois la numérisation comme une déshumanisation du service public, mais malgré cette mise en garde : nous voterons les crédits de cette mission, j'en viens maintenant au crédit de la mission régimes sociaux et de retraite qui font l'objet chaque année d'importants débats relatifs aux régimes spéciaux, je veux avant tout remercier ma collègue Sylvie Vermeillet pour son rapport comme d'ailleurs l'ensemble des rapporteurs spéciaux et pour avis de ces 2 missions, pour ses rapports très éclairant, comme cela a été dit la mission finance principalement le régime de retraite des agents de la SNCF, le régime des marins, le régime des anciens mineurs en Laurent attribuant une subvention d'équilibre nécessaire du fait du déséquilibre démographique, les crédits évolue de manière plutôt stable dans l'ensemble, même si l'examen au cas par cas des régimes révèle des dynamiques variable si les régimes en extinction, c'est logique, hein, mine c'est top voient leurs crédits baisser du fait de démographie en forte baisse, les régimes de la SNCF et de la RATP voient quant à eux, leurs besoins de financement augmenté augmenté assez sensiblement, seul le régime des marins connaît une relative stabilité, le gouvernement a annoncé une réforme des retraites en 2019 mais nous formulons comme souhaité que cette réforme soit enfin celles qui permettent d'assurer définitivement la pérennité de notre système de retraite et de garantir plus de justice entre les cotisants, cette réforme devra conduire à la mise en place d'un système universel de retraite, capable, bien sûr, de prendre en compte les spécificités de chaque métier, la fin des régimes spéciaux ne signifie pas l'égalitarisme, bien sûr, pourquoi certains bénéficieraient de conditions très favorables, quand d'autres doivent travailler des années de plus pour bénéficier de droit parfois moins avantageux ainsi, comme l'a exprimé notre rapporteur pour avis, nous ne pouvons pas accepter que la réforme de l'âge de la retraite votée en 2010 commence à peine à s'appliquer à la SNCF où l'air, le gouvernement a engagé un cycle de discussions avec les partenaires sur sociaux afin de proposer une loi cadre, nous nous donnons donc rendez-vous dans les prochains mois pour aborder cette question qui est au coeur de la vie de nos concitoyens et dans cette attente, mais, chers collègues, notre groupe votera les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole Monsieur Jérôme Durand pour le groupe socialiste pour sa minute. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'attarderai principalement sur la mission Ressources humaines et je veux saluer ici une nouvelle fois le travail de la rapporteure notre collègue Catherine Di Folco malgré nos divergences d'appréciation sur cette mission comme socialistes, nous sommes bien placés pour connaître la difficulté qu'il y a à concilier une politique de ressources humaines ambitieuse dans un contexte budgétaire tendue contexte que traversent nos collectivités territoriales, nos élus ont d'ailleurs accompli des efforts importants sur cette thématique dans nombre de collectivités que nous gérons, nous partageons certains objectifs du comité action publique 2020, 2 installé par le gouvernement, notamment la mise en oeuvre d'un environnement de travail, moderniser, ainsi qu'un souci marqué de simplification, nous craignons toutefois une approche exclusivement comptable qui n'est pas sans rappeler la défunte révision générale des politiques publiques RGPP, par ailleurs, je ne partage pas l'avis de la rapporteur sur le jour de carence tout d'abord, comme le rappelait monsieur Macron quand il était ministre l'inégalité avec le secteur privé est discutable aujourd'hui puisque bon nombre de conventions collectives prennent en charge ce jour de carence, ce qui démontre que son utilité et limitée ou contestables, surtout le récent rapport de l'INSEE est venu nous apporter des éléments tangibles pour discuter l'efficacité de la mesure et si on n'est pas dans l'idéologie et qu'on est pragmatique, on peut observer des faits qui sont indiscutables, certes, la prévalence des absences de 2 jours aurait diminué de plus de 50 en raison de l'application du jour de carence entre 2012 et 2014 et je sais que cela suffit à convaincre plusieurs de nos collègues et de nombreux élus locaux employeurs territoriaux, mais la principale leçon de ce rapport, c'est l'augmentation de 25 pourcent de la prévalence des absences d'une semaine à 3 mois, certains y voient la traduction dans l'esprit de revanche chez les agents notamment territoriaux, la crédibilité de cette hypothèse, m'apparaît fragile et son impact éventuel, certains se félicitent de ce report des absences courtes vers les absences longue, ce n'est pas mon cas, cela facilite peut-être la réorganisation du travail, mais je ne suis pas en mesure de conclure que c'est une bonne nouvelle, ni pour les finances publiques, ni pour la santé des agents publics au-delà de cette épineuse question, nous connaissons les réticences exprimées par les syndicats de la fonction publique sur le report du protocole parcours professionnel carrières et rémunérations le politique PPCR et la compensation prévue pour la hausse de la CSG qui ne permettra pas une hausse du pouvoir d'achat, les collectivités territoriales, attendre d'être pleinement rassuré concernant leurs finances par rapport à la mise en place de cette compensation, enfin, on peut se féliciter de l'augmentation des crédits de formation et de l'effort consenti par l'apprentissage, monsieur Duceppe, Monsieur le Ministre quand vous doutiez encore vous aviez cru utile d'interroger le gouvernement sur la compensation de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité pour les collectivités, le niveau de compensation dépendra de la proportion d'agents bénéficiaire de la suppression de la CES dans leurs effectifs, ainsi la compensation pourra varier selon la répartition des effectifs entre les catégories A, B et C, les collectivités ayant le plus d'agents relevant de la catégorie C seront nécessairement perdante. Pouvez-vous nous garantir la neutralité de l'augmentation de la CSG pour les employeurs, maintenant que vous êtes sûr marche je profite également de votre nouvelle casquette monsieur Duceppe pour interroger le gouvernement sur les salaires versés aux enseignants pour rémunérer les activités périscolaires qui subiront, eux aussi, la hausse de la CSG, comment seront-ils compensés de même les contractuels bénéficieront-t-il une baisse de leur taux de cotisations Urssaf, comme dans le privé, de manière à compenser la hausse de la CSG, vous aurez compris que le groupe socialiste porte un avis pour le moins réservé sur la mission Ressources humaines et choisira par conséquent de voter contre sa mission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. à travers cette mission et au regard du peu de temps imparti, je ne vais pas entamer ici un débat sur les retraites, si la mission de la gestion des finances publiques et des ressources humaines nous donne l'occasion d'évoquer la situation des personnels de l'État et des retraites de la fonction publique d'État, elle nous donne également l'occasion d'évoquer jeudi bien évoquer les régimes spéciaux, ceux-ci obéissent à des règles souvent très complexes, parfois avantageuses et dont les déséquilibres démographiques voire financiers oblige à une intervention de l'État. Nous savons que tous ces régimes sont issus de notre histoire, ils sont antérieurs à la création de la Sécurité sociale en 1945 ils ont été créés pour compenser la pénibilité de certains métiers ou pour répondre à des motivations diverses comme la nécessité de fidéliser un personnel qualifié, ou bien encore la volonté de récompenser ceux qui exercent un métier vital pour la nation. Nous sommes conscients que le meilleur moyen de relever les défis de demain, ce n'est pas dans le statu quo. Si l'universalisation est bel et bien l'objectif, il sera nécessaire de poursuivre la réflexion sur les critères de pénibilité qui devront prendre en contre l'héritage des régimes spéciaux. à l'heure où le haut-commissaire à la réforme des retraites commence à rencontrer les partenaires sociaux, il nous paraît essentiel d'adopter un discours de vérité et de ne pas opposer les différents régimes entre. En effet, faire passer par exemple les cheminots pour les prévenus pour des privilégiés, est une gageure. Les dernières déclarations du gouvernement tendent à proposer une réforme étalé dans le temps afin de ne pas bouleverser les parcours de vie. Cette période de transition pourrait permettre une unification en douceur des régimes, le temps de faire converger les différents taux de cotisation. Ces cotisations ne doivent pas être considéré comme un impôt comme décharge elle constitue en réalité une épargne qui donne droit à un revenu, oserais-je dire universel différée et garanti par l'État. Ce qui nous paraît essentiel, c'est d'assurer la justice et la pérennité de notre système de retraite dans son ensemble. Vous le savez, nous sommes très attachés au système par répartition, il va sans dire que le groupe socialiste sera extrêmement vigilant sur cette question. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics pour 10 minutes. minutes. Le président Monsieur, le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, les crédits de la la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines, la mission Action et transformation publiques les crédits rhénan répartis ainsi que les crédits du compte d'affectation spéciale opérations immobilières de l'État en fait l'objet de 2 rapports spéciaux d'autres commissions des finances par monsieur le sénateur Claude Nogent et Thierry Carcenac, que je remercie pour leurs observations, la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines, les moyens de fonctionnement et d'investissement 2000 des ministères économiques et financiers, les crédits qui sont inscrits financent en particulier le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de l'État, ainsi que les activités douanières les fonctions d'État-Major d'expertise, de conseil et de contrôle, mais aussi les politiques de formation des fonctionnaires d'Action Sociale interministériel et d'apprentissage avec presque 11 milliards d'euros, les crédits de la mission en péril 2018 sont stables par rapport à la loi de finances initiale de 2017 qu'il me soit permis de commencer par les sujets Fonction publique vous rapporteront souligne cette mission contribuer façon importante à la maîtrise des effectifs de la fonction publique d'État, puisque les effectifs du ministère diminueront de 1450 équivalents temps plein en 2018, c'est-à-dire un taux d'effort de 1,1 j'appelle votre attention sur le fait que le ministère de l'action des comptes publics et particulièrement la DG Philippe a beaucoup beaucoup beaucoup contribuer à la réduction du nombre d'agents grâce à un mouvement très important de numérisation, notamment pour le paiement en ligne et qu'il le fait sans sacrifier à ses missions essentielles, notamment grâce au redéploiement des moyens humains là où ceux-ci sont nécessaires, je pense au renforcement des effectifs de la direction générale des douanes et droits indirects, en particulier dans le cas du rétablissement des contrôles induit par le retrait du Royaume-Uni, de l'Union européenne, je souhaite fait il y a rassuré, messieurs les rapporteurs et votre assemblée sur la compatibilité de ses trajectoires des emplois avec la réforme fiscale importante et conduit les services du ministère, la réforme du prélèvement à la source et préparé depuis l'été 2015 en mode projet avec une implication au plus haut niveau et une gouvernance décliner jusqu'aux niveaux les plus opérationnelles la DGF, il se prépare à plusieurs niveaux juridique d'abord tous les textes d'application ont été publiés au niveau informatique aussi le prélèvement à la source a été préparée dès l'été 2016, au niveau de l'accompagnement du changement des agents un correspondant prélèvement à la source, a été nommé dans chaque direction fin 2016, une campagne de formation initiale, s'agissant d'autres réformes comme l'impôt sur la fortune immobilière la taxe habitation ou le prélèvement forfaitaire unique, la DG FIPA et associés en amont aux réflexions et aux travaux, ce qui a permis d'anticiper les travaux informatique et organisationnelle, les éléments de calcul de l'IFI et du pays fut pourront ainsi être déclaré en même temps que les revenus du printemps 2018 et seront prises en compte dans les avis de l'été 2018 : la réforme de la taxe d'habitation sera prise en compte dans les avis qui seront transmises aux usagers à l'Automne 2018 comment analyser en détail vous rapporteur il y a des Philippe et les douanes ont conduit et continuera mais continuent à mener une vaste restructuration de leur réseau territorial avec comme objectif d'accompagner les mutations socio-économique et l'organisation politico-administrative mais aussi de s'assurer que les implantations locales du ministère en bien la taille critique pour offrir un meilleur service aux usagers, aux entreprises et aux collectivités publiques, tous ces projets reposent sur une concertation large avec l'ensemble des interlocuteurs concernés, Philippe à mener des concertations dès l'été, dans chaque territoire avec l'ensemble des élus concernés, avant que les décisions de fermeture de structures ne soit prise par ailleurs la rationalisation du réseau, la réduction du nombre de structures sont systématiquement conçu en fonction de la carte intercommunale, la plupart des fermetures prévues pour 2018 s'effectueront ainsi en fonction du regroupement des EPCI, enfin, nous nous efforçons de trouver des sols conscient concrètes pour assurer toutes les transitions par des permanences au moment clé pour la télé publique, notamment lors des campagnes d'impôt sur le revenu, mais aussi par des permanences régulières au sein des maisons de service public, s'agissant du risque, certains d'entre vous craignez d'affaiblissement du contrôle fiscal, il faut rappeler que l'action de la DG clips sur l'ensemble du territoire en matière de contrôle fiscal participe à l'égalité des citoyens devant l'impôt est assuré indépendamment de l'implantation géographique des services par ailleurs l'examen de de comptabilité qui constitue un nouvel outil au service du contrôle fiscal n'a pas vocation à rencontrer à remplacer les contrôles sur place, mais simplement ouvrir de nouvelles modalités de contrôle à distance et plus rapide, enfin le renforcement du rôle des directions du contrôle fiscal atterrit maître interrégional dans le pilotage du contrôle fiscal répond à la nécessité, disposer d'une vision plus large des problématiques fiscales des entreprises de mutualiser les compétences des agents et de capter les contrôles pratique des contribuables. des DGF, il s'est aussi dotée en 2013, d'un service d'analyse des données pour améliorer la programmation des contrôles fiscaux, avec pour objectif d'être à l'origine d'environ 20 pourcent des contrôles, il est chargé par ailleurs de travaux visant les fraudes des particuliers, dans le prolongement de l'avis de la CNIL du 20 juillet 2017, vous avez été nombreux à souligner, lire les difficultés pour recruter des profils particuliers comme spécialiste en droit, l'immobilier ou des Data scientists ces difficultés sont réelles, pour autant, des possibilités de recrutement spécifique pour les métiers en tension, en particulier dans le numérique existe, et ont été récemment rappelé par une circulaire du 1er ministre le niveau de la rémunération, regardez ce qu'endurent démarche de constituer une difficulté dans administration doit être en mesure développer d'autres facteurs d'attractivité, notamment au regard de l'intérêt des tâches confiées. Je veux aussi rappeler que pour permettre à l'ensemble de ces actions de modernisation et de réorganisation, il faut insister sur le fait que les crédits de fonctionnement du ministère sont maintenus les crédits hors masse salariale s'élève à 2 milliards 175 millions d'euros et progresse de 3,5 pourcent par rapport à l'laquelle les crédits d'investissement qui permettent de conduire les projets informatiques et numériques porteur simplification et de meilleurs services sont aussi en forte hausse de 38 pourcent en matière de transformation, les ministères économiques et financiers sont engagés depuis déjà de nombreuses années dans la dématérialisation des relations entre usagers, administration, chacun peut voir qu'administration fiscale en effet des outils particulièrement performant qui mériterait d'être pris comme modèle dans beaucoup d'action de l'État, cela m'amène à mon second point une nouvelle mission intitulée Action et transformation publiques composé de 2 programmes de 349 et 348 missions qui aura pour objet de transformer durablement l'action publique, je pense en particulier au fond pour la transformation public doté de 200 millions d'euros d'Automne d'autorisations d'engagement 2018 qui modifiera la façon d'envisager les réformes structurelles, l'objectif est d'investir aujourd'hui pour économiser, demain, ces projets devront donc permettre un retour sur investissement, en terme de économies pérenne tant de fonctionnement que 2 visages des investissements se font non pérenne financera donc sur la base d'appel à projets des réformes, générant des économies pérennes et justifiant un surcoût d'investissement transitoire les projets sélectionnés pourront notamment être issue du programme de réformes initiées par le gouvernement programme intitulé Action publique 2022 du travaux du comité d'action publique 20 2022 permettront notamment d'identifier des réformes structurelles, mais aussi des économies significatives et durables sur l'anchois, l'ensemble du Champ des administrations publiques, ils déboucheront sur la mise en oeuvre opérationnelle des plans transformation à partir de 2018 actions publique 2020, 2 pourra aussi compter sur la professionnalisation de la politique immobilière de l'État, ni mission confiée au ministère de l'action et des Comptes publics qui mobilise des moyens financiers du compte d'affectation spéciale opérations immobilières de l'État, doté de 582 millions d'euros avec une hausse de 11 pourcent il faut rappeler que ce compte est un compte spécial qui permet d'affecter les produits de cession des biens immobiliers et depuis 2017 certaines redevances de nature immobilière pour contribuer au financement des politiques avec la avec la proposition de création du programme 348 dédiés à la rénovation des cités administratives et doté d'un milliard d'euros sur le quinquennat marquons notre volonté d'augmenter encore plus la dépenses immobilières consacré à l'investissement et à la responsabilité, en lui confiant la qualité d'être responsable de ce programme, je pense à la direction de l'immobilier d'État je relève avec satisfaction que vous avez bien voulu souligner mesdames et messieurs les sénateurs, les progrès dans la politique immobilière de l'État, avec la création de cette direction, la réforme de la gouvernance matérialisée par la création de la CNIL et la meilleure intégration des outils budgétaires, je vais aussi vous rassurer sur le niveau d'achèvement de la réforme, la charte de gestion a été diffusée l'été dernier, la circulaire sur la pays est en cours d'examen, le devenir des loyers budgétaires a été débattue et continue de faire l'objet de travaux et le dispositif de suivi de la performance et sans cesse améliorer. Je souhaite aussi dire quelques mots dans le temps qui m'est imparti concernant les crédits que l'État consacrera aux pensions de retraite votre commission des finances, a consacré un rapport spécial sur les régimes sociaux à madame la sénatrice et Sylvie Garnier, que je remercie pour ces observations, l'État prend en charge et 55 milliards d'euros, que le régime de retraite des fonctionnaires d'État Bertrand 2018 à ces 2 millions de retraités il verse en outre Sixt virgule 3 milliards d'euros de subvention d'équilibre aux régimes spéciaux de retraite, l'État finance ainsi 20 pourcent des dépenses du système de retraite français, ce qui a souligné. La démarche de transparence du ministère d'action et des Comptes publics vis-à-vis des représentants de la nation se traduit aussi par une document ne augmentation plus riche et qui avait souligné pour les différents régimes de retraite. Sur les différents points qui ont été évoqués et sans pouvoir être exhaustif, du fait du temps imparti, je voudrais simplement dire un dernier mot sur la mission des crédits non répartis vous vous confirmez mesdames et messieurs les rapporteurs que la provision qui avait été inscrit des rémunérations a été répartie lors de l'examen à l'Assemblée nationale sur les titres 2 des différentes missions budgétaires afin de permette l'instauration d'une prime de compensation de la hausse de la CSG, la compensation de la hausse de la CSG pourra plusieurs formes d'abord la suppression de la CES pour les agents publics qui sont assujettis, la provision de 200 99 1000 5 millions d'euros inscrit dans votre finance par l'Assemblée et que nous vous demandons avoir confirmé pour permettre le versement d'une prime de compensation et depuis le 30 ans dans le dernier, le Conseil national d'évaluation des normes a été saisie d'un décret permettant l'abaissement des cotisations employeurs maladie de 11,5 à 9,9 ainsi d'un point de vue macro-économique, l'intégralité des coûts liés à la hausse de la CSG seront compensés les employeurs seront en capacité de consacrer de compenser pour chacun des agents, la hausse de la CSG et en écho Durand et à sa question sur les doutes qui peuvent habiter les uns ou les autres, je voudrais simplement souligner que dans un passé récent, et alors que nous partagions systématiquement les mêmes votes, nous aurions été l'un et l'autre très heureux de voir les coûts salariaux des collectivités et des employeurs territoriaux, notamment pour la mise en des activités périscolaires être compensée de la même sorte je m'arrête là pour la présentation des crédits de la mission et je vous remercie de l'attention, vous avez bien voulu porter à mes propos. Merci monsieur le ministre, donc Les interventions sont terminées, nous allons passer. Sur la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines à l'examen des amendements. 3 amendements, tout d'abord le 233, monsieur le rapporteur pour la commission des finances. Oui, Oui, Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui dirait annuelle habituellement portés par le rapporteur général concernant donc le jour de carence, l'article 48 du présent projet de loi de finances prévoit la restauration d'un jour carence dans la fonction publique, on l'a évoqué, un amendement propose de porter ce délai à 3 jours par mesure d'équité, d'égalité avec les salariés du secteur privé qui sont soumis à ce même délai il tire les conséquences de la modification proposée par le Sénat à l'article 48 l'économie liée à la restauration d'un seul jour de carence élèverait pour la seule fonction publique d'État, à 108 millions d'euros et 270 millions d'euros pour l'ensemble des administrations publiques porter ce délai à 3 jours, se traduira donc par hypothèse, par une économie supplémentaire de l'or de 216 millions d'euros, cette réduction est imputée sur les crédits de la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines d'un souci de clarté des débats parlementaires lisibilité amendements adoptés par la commission des finances. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour la ville et Merci Monsieur le Président, la l'avis du gouvernement est défavorable au fait de porter 2 à 3 jours, le nombre de jours de carence en cas d'arrêt maladie ordinaire pour les agents de la fonction publique, le rétablissement du jour de carence par la loi de finances pour 2018, a été adopté par l'Assemblée nationale et proposé vote d'autres assemblées, nous notons qu'à l'exception des groupes communistes, républicains, citoyens et des groupes France insoumise de l'Assemblée, aucun groupe parlementaire dans aucune des 2 autres, désormais, à l'exception de ces 2 n'ont proposé de revenir sur les dispositions proposées par le gouvernement, nous considérons que le rétablissement d'une journée de carence est suffisant que par ailleurs la comparaison avec la situation des salariés du secteur privé, souffre d'un défaut qui tient au fait que si l'indemnisation par la Sécurité sociale ne prend effet qu'au 4ème jour d'arrêt, certains employeurs complètent le dispositif dans le cas de conventions collectives, la plupart du temps et limite la portée du délai de carence, c'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite maintenant rétablir le jour de carence, comme cela était inscrit dans la loi de finances, mais ne pas aller au-delà d'une journée. Merci monsieur le ministre, j'des demandes d'explications de vote Monsieur Oui, monsieur le rapporteur, présentant cet amendement, nous avait dit : c'est l'amendement habituel que porte le rapporteur général, chaque année, on a vu du soutien à des amendements plus consistant lui mais vous avez raison, d'une certaine façon, vous êtes chargé ce soir de porter vieux marronnier de la majorité sénatoriale, et comme tout vieux marronnier, il faut le traiter comme tels, je pense que c'est une simple provocation et donc il mérite pas sur le fond, après de développement beaucoup plus ample, ce qui serait bien c'est qu'on évite chaque année d'avoir ce type d'amendement, alors c'est vrai, on l'a évité l'année dernière puisque on n'a pas finalement traiter le PLF l'année dernière, c'était donc une année de repos et là on voit revenir les 2 vieux marronnier voilà faisant en sorte que ce soit la dernière année. Merci, cher collègue Madame Cohen pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le le président aujourd'hui elle elle. Contexte de la fonction publique, je l'ai dit, elle est marquée par des années de révision générale de politiques publiques de transfert de charges et d'effectifs, de blocage des promotions et de précarisation des personnels notre collègue du groupe, les républicains nous propose de réduire encore les Budgets en faisant porter à nouveau l'effort sur les fonctionnaires, l'amendement 233 consiste à s'appuyer sur les 216 millions d'euros d'économies dans les dépenses de personnel de l'État, du fait du rétablissement du jour de carence des fonctionnaires en arrêt maladie et de l'allonger à 3 jours en l'alignant sur les salariés du privé tout en omettant de rappeler que pour les 2 tiers des salariés, l'entreprise prend en charge les 3 jours de carence et je vais parler aussi de l'amendement 230 parce que c'est dans la même logique, lui, part de l'idée selon laquelle les fonctionnaires ne travaillant pas autant que les salariés du privé, il conviendrait de ramener le temps de travail effectif des agents du service public de 35 à 37 heures 30 ce qui permettrait évidemment de réaliser une économie de 2,2 milliards d'euros, la logique de notre collègue nous et donc le traitement des fonctionnaires dont le point lundi, dont le point d'indice et je l'ai pratiquement depuis 2010 ne connaissent non seulement aucune progression mais encore soit affectée par 2 jours de carence supplémentaire et par 2 heures 30 hebdomadaire de travail supplémentaires non rémunérées fonctionnaires travailler plus et gagner moins, telle est la philosophie de ces 2 amendements que nous ne pouvons partager et c'est pourquoi nous voterons contre les 2 et pour une fois, je dirais, une fois n'est pas coutume de saumon en accord avec la le le gouvernement souligne. Merci. Alors Madame Katell pour explication de vote. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais, chers collègues, je dirais à notre éminent collègue Claude Reynaert, que je ne porte pas les marronniers d'une majorité sénatoriale et qu'une façon de ne plus parler de marronniers, c'est de voter une disposition au-delà de de de ce très aimable à destination de Claude rénal, je voudrais dire que il ne s'agit pas ici de caricaturer la fonction publique et au travers de cet amendement de considérer que les fonctionnaires ne travailleraient pas assez, je crois que chacun d'entre nous, quand il a géré une collectivité reconnaît la capacité et le sang aiguë du service public des fonctionnaires, je dis juste que il n'est pas tout à fait vrai de dire que l'ensemble des entreprises privées compensent les jours de carence et que moi je pense qu'il y a un critère d'équité, je dirais qu'il n'est pas fait d'aucun mépris au dos d'aucune discrimination à l'égard des fonctionnaires et que je trouve que par équité, moi je suis assez favorable à cet amendement, maintenant je comprends Monsieur le Ministre, que vous ayez décidé de marcher doucement sur ce sujet, je l'entends bien et c'est un avis personnel que j'exprimais. Merci monsieur cadré pour explication d'. monsieur le président, Monsieur le Ministre, effectivement, c'est un sujet que certains qualifieront de marronniers comme vient de le dire Françoise Cathala l'instant il est légitime quand même de réinstaurer ce jour de carence, tout simplement parce que il existait auparavant et puis on a jamais compris pourquoi Madame Lebranchu a absolument voulu le supprimer, tant il est vrai qu'il avait démontré tout à fait son intérêt, puisque l'est analyse ont clairement démontré que l'absentéisme dans les collectivités publiques dans l'ensemble de la fonction publique avait significativement diminué au moment où ce jour de carence fut instaurée et donc de ne pas le institué serait eux totalement normal, pour des raisons d'équité combien encore de le dire, notre collègue Françoise Katell c'est absolument légitime que ceci soit soit instauré en tout cas on ne peut pas comprendre mais on ne peut pas demander au à l'ensemble de la fonction publique, de gérer les ressources humaines, sans avoir les outils pour cela. Merci monsieur le ministre. le monsieur le président, il ne s'agit pas pour moi de de rassurer Madame Katell sur le rythme de ma marche, mais simplement d'apporter une précision, en écho aux propos de Madame la sénatrice, quand même, vous avez eu raison de rappeler, madame, que le point d'indice avait été de 2010 à 2016 et le jet d'un dégel 2 fois 0,6 points en 2016 avec une application 2017, par contre, le propos, vous avez des mots apporter une précision au type de l'année 2017 la reconduction du gel du point d'indice pendant les 6 années j'ai évoqué, comme en 2018 ne sera du pas nécessairement par une stagnation totale de la rémunération des fonctionnaires puisque sur l'année 2017 l'application avec le décalage de 6 mois, de ces 2 légère revalorisation du point d'indice, l'application d'un certain nombre de mesures catégorielles et la mise en oeuvre des premiers éléments du PPCR pour les années 2016 et de 17 ont amené la rémunération mensuelle moyenne des agents publics a augmenté de 4 pourcent ce qui est un niveau d'évolution qui est largement supérieure à l'intégralité des années précédentes et je pense aux 10 ou 15 années précédentes, donc il y a une progression tout le monde peut souhaiter qu'elle soit plus forte, évidemment, mais il y a une progression de la rémunération en tout cas de la capacité des fonctionnaires dans leur pouvoir d'achat progressait indépendamment des seules questions d'indices mais liés aux mesures catégorielles au PC. Merci, monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai été saisi d'une demande. C'est un public par le groupe CRC sur l'amendement 233 de la commission des finances, je vous rappelle que l'avis du gouvernement a défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 39 sur l'amendement 230 2 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs du groupe politique et notifié à la présidence, le nombre de votants 330 nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 189 contre 140 le Sénat a adopté. Nous poursuivons l'examen des amendements avec le legs de l'amendement 230 de la commission des finances, monsieur le rapporteur.

dans son enquête sur la masse salariale de l'État a réalisé en 2015 la Cour des comptes estimait qu'une augmentation de 1 pourcent du temps de travail, la fonction publique se traduirait par une économie de 700 millions d'euros pour l'ensemble de la fonction publique. C'est-à-dire 5,4 millions d'agents, l'aliment de la durée du travail d'un secteur public sur le temps de travail habituel en secteur privé permettrait par conséquent un gain de 5 milliards d'euros rapportés à la seule fonction publique de l'État, c'est-à-dire 2 4 millions d'agents, cette économiste élèverait à 2 2 milliards d'euros, c'est l'objet de cet amendement qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique d'État. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, pour avis du gouvernement. monsieur le président, monsieur le rapporteur ne pardonnera mais cette n'avoir à nouveau un avis défavorable à cet amendement sur différents aspects sur le plan formel d'abord il fait porter au seul programme 156 sur la DG Philippe une économie d'un montant considérable calculé pour l'ensemble du périmètre de l'État, la masse salariale de la direction générale des finances publiques serait alors si cet amendement était adopté, amputée de 32 pourcent et cela aurait pour conséquence un risque évident d'un soutenabilité de la mesure, vous indiquez dans l'exposé des motifs que les économies correspondantes devront être répartis sur l'ensemble des missions du budget général cela méconnaît malheureusement le fait que la répartition des crédits votés par le Parlement au niveau de chaque programme ne peut être modifiée qu'à la marge et sous des conditions précises qui sont encadrées par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et notamment par son article 12 sur le fond, par ailleurs, nous ne souscrivons pas votre analyse un rapport de la Cour des comptes de 2015, qui s'appuie sur les chiffres de l'enquête emploi dès 2012 révèlent que la durée hebdomadaire dans la fonction publique d'État est légèrement supérieure à celle du secteur privé, les économies, vous proposez suppose plusieurs dizaines de milliers de suppressions de postes supplémentaires qui ferait peser par ailleurs un risque de rupture de la continuité du service public au sein des administrations de l'État, j'ajoute que nous avons initié, je l'évoquais tout à l'heure, en réponse à certaines interrogations, le programme avec son public 2020 avec un comité d'experts 4 22 avec 5 chantiers transversaux qui sont portés par les différents ministères avec 13, forme de l'action publique et avec la mise en place actuellement d'un comité de suivi association et associant les organisations syndicales, l'objectif est de proposer des pistes de transformation et de modernisation de l'action publique des pistes de réforme et de modernisation des administrations qui nous permettrait de pouvoir rendre le même service, la même qualité de service tout on n'interrogeant le niveau des effectifs, c'est une méthode de concertation, une méthode de concertation préalables qui serait contradictoire

Merci, mes chers collègues, si vous pouvez être un tout petit peu plus attentif. Et moins bruyant dans l'hémicycle, ce serait bien monsieur presque question de vote. Oui, j'ai pas reprendre le même argument d'autant plus que le le le dossier certes toujours quelque chose, un amendement que l'on connaît, que l'on a déjà vu dans les années précédentes, mais je trouve surtout que donc sur le fondement, je crois que le ministre a répondu sur le temps de travail, il faut être extrêmement prudent sur ces sujets, mais on a tous, on est tous ici dans l'ancien responsable de collectivité territoriale, je sais bien que l'amendement s'applique à la fonction publique d'État et n'est pas la fonction publique territoriale, mais on peut imaginer qu'il ne se passe de translation qui se fait sur les 2, tous ceux qui ont géré des collectivités territoriales, savent que la question du temps de travail n'est jamais posée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a tous en tête des agents de la fonction publique territoriale, en particulier pour ceux qui gèrent et qui faisait très largement plus que leurs horaires sur le papier, on a tout ça en tête, lorsque vous avez un pépin dans une commune inondations etc vous appeler tout le monde arrive et personne de demandeurs supplémentaires jamais vu ça, moi en tout cas non je je trouve que c'est très maladroit, très maladroit de ramener ça à un montant à des principes et ses principes d'ailleurs ne sont pas toujours vrai par contre ce qui est vrai c'est que si on gère mal sa fonction publique, alors si ce n'est pas capable d'avoir un management un peu positif, un peu de travail en commun avec les agents, hé bien c'est vrai, on peut avoir des positions qui sont des positions de retrait et de recul sur le strict minimum, mais c'est à nous tous, finalement dans notre management de trouver les conditions d'un travail en commun qui soit un travail positif et dans lequel les agents soient heureuse de travailler dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d'État, c'est autour de ces sujets-là, je pense qu'on devrait s'investir et pas sur des visions comptables qui se ce roman n'ont pas leur place ici dans cet hémicycle. Merci, cher collègue Madame Cohen pour explication de vote. Oui, très brièvement, parce que notre collègue Reynal a vraiment exprimer ce que je voulais dire, si ce n'est que, effectivement, la façon dont le rapporteur a présenté cet amendement comme le précédent est quand même très désincarnées et que ne se base que sur une une gestion comptable qui ne correspond pas à la réalité des conditions de travail et puis puisque j'ai pris la parole samedi permet de de faire une petite précision par rapport à tout à l'heure si j'étais d'accord avec l'expression du du ministre disant qu'il voulait pas étendre un jour à 3 jours, il est bien entendu qu'on n'a pas changé de position au niveau du groupe communiste, on est absolument opposé au jour de carence qui en est à un, 2 ou 3, voire plus, mais je le dis parce que ça pourrait entraîner une ambiguïté à cette heure tardive, et comme tous mes collègues étaient attentifs, je reprécise les choses. Merci, cher collègue, donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public, parce le groupe CRC. Pardon Madame espoir si ça sonne pour explications de vote. Non, Monsieur le Président pour demander une suspension de séance de 5 minutes. Oui vraiment 5 minutes maximum, merci, je le leur ai déjà avancé, on a notre mission derrière, donc c'est 5 minutes maximum. Merci beaucoup. Et

La séance est reprise. Donc, sur l'amendement 232 de la commission des finances, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC, je vous rappelle que l'avis du gouvernement défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

Mais, chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 39 sur l'amendement 230 2 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs du groupe politique et notifié à la présidence, le nombre de votants 330 nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 189 contre 140 le Sénat a adopté. Nous poursuivons l'examen des amendements avec le 231 monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, bon tout à l'heure j'ai indiqué la révolution numérique touche bien évidemment les administrations de réseaux que sont la DGF Philippe et les douanes, recruté en tant que contractuel, une vingtaine de tonnes ça scientiste et de Data analyste disposant d'un niveau de compétence en matière d'analyse l'exploitation de données de masse paraît essentiel ses compétences sont aujourd'hui devenues cruciales, en particulier le recours à des algorithmes prédictifs permettrait un meilleur ciblage des risques et puis une meilleure identification des âges et infinie, un meilleur service public, notamment dans la lutte contre la fraude fiscale Panama pêche percé par Papers l'ont démontré, or l'administration éprouve des difficultés à recruter et fidéliser ces profils atypiques, le présent amendement vise à apporter une meilleure réponse, c'est un amendement d'appel également permettant le recrutement de, de, d'une vingtaine de Data scientists si on compare les rémunérations dans le privé, on se rend compte que c'est essentiel, monsieur le ministre, vous avez rappelé tout à l'heure dans votre propos que la circulaire du 1er ministre permettez et ouvrait des possibilités de de recrutement, or on se rend compte que, dans les fêtes il n'allait pas ainsi, c'est en ce sens que la commission adoptées se présente un amendement qui a pour effet de de faire basculer un 1000000 4 d'euros et permettant de de pouvoir recruter ce type de personnel. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour la vie et gouvernement. Merci monsieur le président, et merci au rapporteur Thierry Carcenac de cet amendement, j'ai entendu, c'est un amendement d'appel et qui permet de mettent l'accent sur à la fois l'impact des nouvelles technologies sur les métiers du contrôle, notamment au sein de des j'flippé, le DG des délits et d'autre part de l'attractivité des métiers numérique au sein de l'État, de la capacité de l'État à recruter des profils, au niveau de compétence, j'ai effectivement signalé tout à l'heure qu'une circulaire permettait d'ajuster un certain nombre de choses et que d'ailleurs, l'État avait recruté une vingtaine de l'hôtel, en ce qui concerne l'exploitation des données de masse la DGF IP DG DDI sont déjà pleinement engagés dans une démarche qui vise à renforcer, au moins au moyen d'outils numériques performants, la perfide la paire faut que la pertinence pardon et l'efficacité du ciblage des contrôles et nous sommes ainsi dotés en 2013, un service d'analyse de données pour améliorer la programmation des contrôles fiscaux, ce service chargé initialement d'expérimenter de nouvelles techniques et méthodes d'analyse devra partir 2018 s'intégrer de façon tout à fait opérationnel, donc dans la programmation du contrôle fiscal des professionnels avec pour objectif d'être à l'origine d'environ 20 pourcent des il est chargé par ailleurs des travaux visant la fraude des particuliers, dans le prolongement de l'avis de la CNIL 20 juillet 2017 que j'ai évoquée tout à l'heure, cette montée en puissance du service nécessite encore certains investissements humains et matériels dans la rénovation de l'intégralité de l'architecture informatique sur laquelle sont réalisés les analyses le travail d'appropriation développement informatique des travaux de programmation réalisés actuellement dans les services déconcentrés et l'acquisition éventuelle de logiciels d'analyse dans les données textuelles ou de robots d'Intelligence artificielle pour exploiter des données plus massif d'origines diverses, notamment des données extraites d'Internet en ce qui concerne la direction générale des douanes arrêté du 29 février 2016 crée le service à compétence nationale dénommé service d'analyse de risques le ciblage qui est en charge de la production des analyses de risques et les études à vocation opérationnelle pour le dédouanement et la fiscalité, il développe notamment les techniques de Dataminr afin de repérer les schémas de Freud atypique, le DG Philippe et la Direction des douanes sont donc déjà dotée de moyens technologiques budgétaires et humains destinés à renforcer la pertinence et l'efficacité de leur contrôle des investissements tant humains que matériels doivent encore être réalisés en 2018, mais il n'apparaît pas pertinent, comme le propose l'amendement s'il était adopté, de les effectuer au détriment de la Snecma salariale du programme de 78 dans certains services, tels que Tracfin lutte également contre la fraude fiscale, par ailleurs, j'ajoute que dans le cas du grand plan investissement 300 millions d'euros par an ont été flashé sur les questions de formation afin d'développer les compétences d'accompagner les transformations de former aussi les agents publics à l'exercice de nouveaux métiers que par la formation des agents présents dans nos services des directions de l'État souhaite aussi se doter de moyens humains en capacité de répondre à vos préoccupations, c'est la raison pour laquelle je suggère, monsieur le rapporteur, puisse se retirer votre vraiment il y a des faux ça sera vie favorable. Merci monsieur le ministre, oui, monsieur le rapporteur. Oui monsieur pertinent, merci monsieur le ministre, c'est un amendement d'appel puisque vous l'avez bien noté cette difficulté de de recruter existe, même si vous nous avez indiqué qu'il y a effectivement des personnels qui sont recrutés, compte tenu des difficultés de rémunération par rapport au privé, les personnes ne reste pas forcément, et nous avons de très grosses difficultés dans nos services, ça a été indiqué par les directeurs généraux et nous étions avec monsieur Mougin et moi-même, dans le cadre de ses positions et puis nous avons rencontré également le directeur de la dynamique est également, c'est un point qui est soulevée, donc je vous remercie de la réponse que vous nous avez apporté mais j'aurais l'occasion avec l'amendement suivant de revenir sur ce sujet donc je retire l'amendement. Merci monsieur rapporteur amendement est retiré, donc je vais mettre aux voix, les crédits de la mission. Gestion des finances publiques et des ressources humaines qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. Je mais au Boilard le 55 terre qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté après la. 55 terre un amendement 230 rectifier, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, bien cet amendement vient dans la suite de ce que j'ai indiqué notamment sur la difficulté de à recruter et puisque vous avez indiqué que nous avions toutes les capacités pour pouvoir recruter un rapport sur l'opportunité de créer un indicateur de performance de la mission en gestion des finances publiques et des ressources humaines, rendant compte de l'attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d'information et de la communication, son état serait les bienvenu, c'est le sens du c'est le sens Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, la Direction interministérielle du numérique et du site du système d'information de communication de l'État, placé sous l'autorité du 1er ministre et qui pilotent avec la direction générale de l'administration de la fonction publique, le plan d'action permettant d'attirer, de recruter et de fidéliser les compétences rares nécessaires à la transformation numérique de la science de l'action publique, comme le rappelle la circulaire du 1er ministre du 21 mars 2017 travaille à améliorer les conditions de l'attractivité de la filière des métiers du numérique au sein de l'État, il y a de nombreux groupes de travail qui sont en cours sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs des compétences sur les rémunérations sur le recrutement sur la mobilité, ainsi que sur les formations dans les métiers du numérique comme je l'évoquais il y a un instant dans les services, toujours de l'État, l'ensemble de ces groupes d'être de travail devraient aboutir au cours de l'année 2018 aussi, nous sommes prématuré, lancer une mission sur ce thème, car nous préférons très simplement consacrer les efforts des Serbes, des services à l'aboutissement de ces travaux qui déboucheront très prochainement, et donc non pas que nous ne souhaitions pas rendre public ou produire un rapport sur cette question de l'attractivité nous considérons par contre qu'il serait plus efficace de se réunir et de faire ensemble un bilan à l'issue des groupes de travail, c'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable, si vous me permettez, Monsieur le Président, simplement pour pour s'il que de manière assez générale, nous soulignons et nous rappelons que plutôt que des rapports gouvernementaux, nous suggérons ainsi qu'aux parlementaires de se saisir leur Gatti dans le cadre des exercices de contrôle et de mission d'information.

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Je mais au mois les crédits de la mission crédit non réparer. C'est lui Qui est contre. Qui s'abstient qui seront adoptées. Les crédits de la mission Action et transformation publiques même vote. Même vote pour la gestion du Patrimoine immobilier de l'État. Même vote pour les régimes sociaux et de retraite. Et même vote pour le compte spécial pensions. Donc tous ces crédits sont adoptés, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, vous avez indiqué, il y a un instant que d'autres missions budgétaires attendez d'être examinée par votre assemblée la mission suivante et porté par ma collègue, secrétaire d'État, madame Gény-Stephann, qui est actuellement au banc à l'Assemblée nationale, c'est la raison pour laquelle afin qu'elle puisse être présenté, répondre aux questions de votre assemblée, je sollicite au nom du gouvernement une suspension de séance de 15 minutes pour permettre que techniquement j'ai puisse la remplacer à l'Assemblée nationale et qu'elles puissent vous rejoindre. Ben écoutez, monsieur le ministre, c'est vrai que c'est pas très apprécié, mais surtout à cette heure tardive, j'avoue que, voilà le Sénat passe après l'Assemblée, si j'ai bien compris

La séance est reprise. J'ai une demande de rappel règlement Madame Prima. Merci monsieur le Président, Madame la ministre, je voudrais à cette heure tardive de la nuit, vous faire un rappel au règlement, le ministre précédent qui était sur ces bancs, est partie précipitamment à l'Assemblée nationale pour vous remplacer, vous arrivez, je vois que vous êtes essoufflé et donc ce n'est pas personnel, mais il existe 4 ministres qui s'occupe de cette mission, nous avons un ministre en charge des relations avec le Parlement, ce qui vient de se passer est juste inadmissible, c'était une demi-heure que nous attendons dans dans le dans l'hémicycle pour parler de la dette de la France, qui n'est pas le plus petit sujet de ce projet de loi de finances, voilà, nous sommes très remonté et je peux vous dire que véritablement, il s'agit d'un incident de séance. Merci. Nous prenons acte de ce rappel au règlement. Qui sera transmis au président. Manille a-t-elle. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais, chers collègues, je vais aussi faire un rappel au règlement, ma société aux propos de notre collègue Sophie Primas Madame la mine sommes heureux de vous accueillir à cette heure tardive au Sénat voulu être strictement pour rien et ne prenait pas mon propos, comme un propos personnel mais je pense qu'effectivement, le Sénat américain de du respect de la considération la dette de la France, encore un peu plus et nous ne pouvons que regretter le fait que les sénateurs étaient abandonnés, comme la dette de la France pendant une demi-heure, c'est fort regrettable. alors nous, nous allons examiner les crédits de la mission engagement financier de l'État, les comptes spéciaux, participation de la France au désendettement de la Grèce participation financière de l'État accords monétaires internationaux et avance à divers services de l'État ou organismes gérant du service public, ainsi que l'émission Investissements d'avenir et remboursements et dégrèvements. La parole est à madame Nathalie Goulet, rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le président de la commission dès les finances, mes chers collègues, la messieurs engagement financier de l'État recours essentiellement les crédits alloués simplement de la charge de la dette 99 pourcent des crédits dans je suis rapporteur d'avant, je voudrais saluer la démarche de nos collègues députés Bénédicte Peyrol Dominique David Kimouyou associé à l'Assemblée nationale à leurs travaux, ce qui est assez inédit et qui était plutôt agréable en 2017, les pays de l'OCDE ont emprunté 9200 milliards de dollars, la faiblesse des taux d'intérêt ont conduit une fois de plus à ce que la charge de la dette diminue, alors même que notre endettement continue à progresser cette situation faussement rassurante ne doit pas nous leurrer la hausse des taux d'intérêt est inéluctable, il faut s'y préparer, d'après l'Agence France Trésor, une hausse d'un point des taux d'intérêt en 2018 nous coûterait 14 milliards d'euros en 2024 et serait absolument insoutenable pour nos finances publiques, cette hausse a commencé en 2017 pour la première fois en 6 ans, nous devons rouvrir les crédits en cours d'année, pour payer la charge de la dette, notre situation est d'autant plus préoccupante que notre niveau d'endettement est très élevé, que les programmes de financement des années à venir, particulièrement lourd, par ailleurs, le montant amortir concernant les dettes à moyen et long terme, vous avez bien fait de rester parce que vous allez pouvoir ajouter ajouter passerait de 127,6 milliards d'euros à 140,3 milliards d'euros entre 2017 et 2018 soit une rose de 10 les amortissements progresse en raison de l'arrivée à échéance des volumes des dettes importants émis lors de la crise économique des années 2000, il s'agit d'un point de tension supplémentaire sur le programme de financement le niveau de la dette publique française est un problème évident c'est aussi un problème pour l'Europe puisque nous ne respectant pas évidemment les critères de Maastricht, vous comprendrez bien, Madame le Ministre, que vous méritez, nous méritons et cette mission mériterait mieux que 10 minutes à minuit le soir dans cet hémicycle, bref au rythme annoncé de désendettement, il faudra 40 ans pour rattraper l'Allemagne donc plusieurs pistes pour un remboursement parce que personne n'en parle mais il va bien falloir un jour diminuer sa dette et la rembourser un ou plusieurs fonds sectoriels abondé par les fonds des États-membres qui refinance serait certaines dates de façon mutualisée, c'est l'idée que défend Thierry Breton avec les fonds spécialisés, notamment pour la défense, la 2ème piste et la création d'emprunt mutualisé de la zone Euro mais ça nos amis allemands ne sont pas tellement favorable 3ème piste la participation du mécanisme européen de stabilité au paiement des intérêts des dettes des États les plus fortement endettés en contrepartie d'un engagement durable et crédits dans un processus de redressement mais enfin de toute façon, il vaut mieux de voir que pas pouvoir rentrer pour l'instant, on promet son pouvoir tenir aucun toutes ces règles conduisent à renforcer l'interdépendance entre les émetteurs de la dette souveraine et les banques, il faut réfléchir à des évolutions possibles, il ne reste pas beaucoup de temps, le sujet est technique, les enjeux colossaux, nous sommes tous fatigués, vous venez d'arriver : donc je vais vous proposer quelques questions auxquelles j'aimerais quand même que vous puissiez répondre parce qu'encore une fois, on est sur 1750 milliards d'euros, on est quand même sur le point, et le budget le plus important de l'État, on traite franchement par-dessus la jambe, donc pourquoi la mission ne pourrait-elle pas Madame le Ministre, faire l'objet de plafond limitatif et non évaluées, que pensez-vous des mesures de désendettement qui pourraient être mises en oeuvre au niveau européen et concernant le traitement prudentiel, parce qu'il va aussi falloir prendre des garanties concernant le traitement prudentiel de la dette souveraine, quelles sont les pistes qui devraient être privilégiée, je voudrais ajouter puisqu'il nous reste une minute que nous avons auditionné longuement les agences de notation et que l'ensemble de nos politiques publiques l'ensemble des promesses que nous faisons et notamment les promesses en matière d'emploi sont scrutés de façon à pouvoir, n'ai pas tout à fait fini de me laisser parler, donc je vous disais, Madame le Ministre, que les promesses qui ne sont pas tenus pénalise notre pays donc j'ai soulevé 3 questions, j'aimerais bien le ministre dans le cas de votre exposé vous puissiez nous y répondons donc je vous indique aussi que la commission des finances propose adopté les crédits de la mission engagement financier de l'État et des comptes spéciaux qui sont associés, j'aimerais aussi que dans le cadre de l'organisation de nos travaux l'année prochaine, nous puissions avoir un peu plus de temps pour débattre de façon éclairée et un peu moins soporifiques de ce poste extrêmement important,

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des finances. De Monsieur messieurs, chers collègues. La commission des finances est réuni sur ce compte d'affectation spéciale. A émis un avis assez inédit. On a décidé de s'en remettre à la sagesse de du Sénat et donc on compte sur le gouvernement pour nous éclairer sur ce qu'on peut d'affectation spéciale participation financière de l'État.

sa participation de l'État à peu près 15 milliards à la BPI et le reste 25 milliards à la CDC, vous savez l'économie générale de ce compte, il doit être présenté en équilibre en général depuis de longues années, sauf l'an dernier, bien écriture conventionnel, une programmation conventionnel dans l'espace, la c'est 5 milliards 5 milliards et qu'en aucun cas il ne peut être déficitaire, le solde annuel cumulé doit être positif. J'avoue que l'exercice qui nous a demandé peut s'apparenter à un exercice de Style. On nous demande de donner l'autorisation selon rôle du Parlement. Ensuite, le gouvernement, c'est ce qu'il veut. Dans pouvoir totalement discrétionnaire et libéré, si j'ose dire, des contraintes de la loi organique. Il nous faut nous parlementaires. Attendre la loi de règlement, donc 6 mois après l'adoption de la LFI pour voir ce que l'État a fait de l'autorisation qui lui a été délivré en fait nous avons presque tous dit et on a voté à l'unanimité, à s'en remettre à la sagesse de cette assemblée, c'est un véritable blanc-seing qui est délivré à l'État. Autorisation sollicitées du Parlement normal obligatoire et un véritable blanc-seing délivré au ouverte. Avec d'ailleurs que peu de contraintes, citons : on regarde bien, il y a quelque temps, en janvier 2014, le gouvernement d'alors avait décidé de s'assigner si j'ose dire, une doctrine d'intervention, d'avoir une philosophie de l'aide de l'État interventionniste de l'État stratège depuis lors, les choses ont beaucoup évolué et on a bien l'impression qu'il y a plus de doctrine et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé sur c'est ce qui s'est passé sur Alstom, 2 philosophies différentes, et si j'ose dire, contradictoire et donc on aimerait bien donc, comprendre ce qui se passe par ailleurs, l'État nous a dit très clairement dans les documents que nous avons tous reçu que il faut financer l'innovation et ovation et déjà par ailleurs financé sur le programme 192 sur la part la CDC et que sais je, bref, il y a un foisonnement de programmes d'actions pour financer l'action apparemment l'innovation apparemment dite de rupture, apparemment ce n'est pas suffisant donc il vous faut 10 milliards placés à intérêt qui devrait rapporter entre 200 et 300 millions désormais se font depuis l'avis émis par la commission des finances a évolué, ce n'est plus fonds d'innovation, c'est un fonds pour l'industrie. Et l'innovation donc politique industrielle et politique d'intervention de l'État et de gestion du Patrimoine de l'État, donc ça demande quelques précisions le 1er ministre a bien voulu. émettent quelques lueurs nous donner quelques éclairages le 20 novembre dernier dans un discours prononcé au Conseil national de l'industrie en disant que tout est stratégique et quand même le yaourt et stratégique et donc il y a des filières qui sont stratégiques, il y a aussi des produits qui le serait-il il y a aussi, c'est la belle marque France hé bien l'État interviendrait donc on a impression que dans la doctrine d'intervention, la communication qui a été faite en janvier 2014 où on disait on va se recentrer l'État régalien va se recentrer sur le souverain le régalien, la défense, la sécurité, maintenant ça peut-être pourquoi dans dans l'agroalimentaire et et dans quelques produits, donc on aimerait avoir quelques lumières surchauffe font pour l'industrie et pour l'innovation, par ailleurs, on aimerait aussi que le gouvernement nous explique comment faire 10 milliards alors désormais, ce sera plus 10 milliards, ce sera 2 milliards qui sera placé pour apporter 200 millions immédiatement

ou peut-être modifier la loi organique pour que les dividendes en nature selon leur nature, pardon, soit en numéraire qui alimentent le budget de l'État, le budget général, soit en titre qui est géré par la paix, il y a là quelques étrangetés que nous aimerions voir éclaircies ce soir donc, on compte sur les lumières du gouvernement pour permettre à l'Assemblée de statut. essayer de ne pas dépasser, si on veut pas se coucher trop tard. Voilà, alors Madame Lavarde, rapporteur spécial, la commission des finances pour 5 minutes. Madame le Ministre, mes chers collègues, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc, vu comme ça, il semble normal que le Sénat parle des investissements d'avenir, à des heures les plus matinal, cette mission a été institué dans le cadre de la loi de finances pour 2017 afin de faire figurer l'enveloppe budgétaire consacrée au 3ème programme d'investissements d'avenir ou pays à 3, soit 10 milliards d'autorisation d'engagement qui s'ajoute aux 47 milliards des 2 programmes précédents initiée en 2010 et en 2014, la mission avait la particularité, en 2017 de bénéficier uniquement d'autorisations d'engagement sans aucun crédit de paiement cette astuce de budgétisation notamment mis en exergue par Albéric de Montgolfier, alors rapporteur spécial de la mission permettait d'éviter que le pays à 3 ne pèse sur le déficit budgétaire dès 2017 l'avenir du pays à trois pouvait apparaître un certain l'été mais son intégration dans le grand plan d'investissement ou j'ai payé le conforte en effet le pays à trois représente 10 des 57 milliards du GP pays cependant on notera que l'effort financier est reporté sur la fin du quinquennat en effet pour 2018 seuls 1,0 8 milliards d'euros de crédit paiement sont inscrits 4 milliards d'euros sur le triennal 2018, 2020, il reste donc 6 milliards à financer au-delà l'inscription de crédits de paiement et tant mieux pour autant leur rythme de décaissements et leur nature, ne peuvent que susciter quelques inquiétudes tout d'abord la trajectoire des décaissements et réalisé en cohérence avec les perspectives globales des finances publiques, ce n'est donc pas le rythme d'avancement des actions du pays a qui détermine l'inscription de crédit mais la simple contrainte budgétaire, il y a là une véritable rupture par rapport aux pays a un et 2, et la gestion des crédits par les opérateurs et de ce fait, rendu plus complexe ce en second les crédits inscrits en 2018 correspondent pour une large part à des prises de participation, fonds propres qui représente l'Avantage certain de ne pas avoir d'impact sur le déficit maastrichtien au contraire des autres modes d'intervention du pays ainsi les fonds propres représentent 70 pourcent de l'enveloppe de crédits pour 2018 et un tiers seulement des avances remboursables, subventions et dotations décennale seront disponibles sur le triennal 2018, 2020 certains opérateurs s'interrogent et nous avec, sur la possibilité de trouver suffisamment de projets à financer par fonds propres, ce risque est d'autant plus, pas tant que l'enveloppe du pays a n'intègre pas de soutien aux dépenses d'ingénieurs et pendant la phase de définition des projets. sur la forme, l'intégration dans le GP il n'a en rien modifié la structure du pays a les programmes et les actions financées la répartition des autorisations d'engagement, la répartition entre les différents modes de financements, les opérateurs chargés de la mise en oeuvre demeure les critiques émises en 2017 par le Sénat demeure donc également le recours à un sous-opérateur doit être circonscrit, car il est source de complexité pour les porteurs de projets et risque de dédoubler les activités d'opérateur, alors même que la Caisse dès que les pays à mobilise déjà près de 180 agents à la Caisse des dépôts et consignations, le versement des crédits aux opérateurs ainsi que les décaissements de ces derniers vers les bénéficiaires continuent à ne pas intégrer être intégrés dans la norme de dépenses, contrairement à la recommandation de la Cour des comptes dans son rapport public de décembre 2015 enfin, le risque pour le gouvernement de procéder à des des budgétisation reste également important sur le fond, certaines actions s'inscrivent dans les axes définis par le gouvernement, notamment toutes celles relatives à la qualification de la main-d'oeuvre à l'innovation, à la transition écologique le coup d'arrêt brutal à quelques jours de la remise des offres de l'appel à projets nouveaux instituts hospitalo-universitaires, illustre la volonté du gouvernement de revoir certaines orientations s'il peut se comprendre que le gouvernement souhaite redéfinir certaines actions en fonction de ses priorités, il convient toutefois d'éviter que les appels à projets histoire subitement stoppée ou des projets essentiels remis en cause, interrogé par la commission des finances, le ministre de l'éducation n'a pas été en mesure de décrire le contenu du nouveau plan numérique à l'école, porté par l'action cette du programme 421 enfin nous moquons pas nous interroger sur le contenu de l'action 9 grands défis du programme 423 accélération de la modernisation des entreprises, ces atermoiements explique certainement le retard pris dans la signature des conventions entre les États et les opérateurs, puisqu'à ce jour, seuls 8 dès 8 conventions attendus sont signés si nous partageons tous l'objectif de maîtrise globale des dépenses publiques, il nous semble qu'utiliser les pays à comme variable d'ajustement, en créant une dose sur Sion forte entre autorisations d'engagement, les crédits de paiement risque d'annihiler tous les effets positifs de cet outil spécifique, pourtant le pays apportent des projets utiles pour l'investissement de notre pays, j'invite donc, ce soir, ce matin, le Sénat a voté les crédits inscrits pour cette année, tout en vous indiquant : Madame le Ministre, que nous serons très vigilants sur leur utilisation. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pascal Savoldelli, rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame et même la ministre chars collègues. La mission remboursements et dégrèvements représente 115,2 milliards d'euros de crédit, soit le montant le plus important atteint depuis que cette mission existe, cela en fait la plus importante mission du budget de l'État, en hausse de 6 pourcent par rapport à l'évaluation 2017 réviser cette hausse significative c'est speak notamment par l'augmentation des dépenses au titre du du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE et des crédits d'impôt sur le revenu et s'agissant des impôts locaux, par la mise en place de la première tranche du dégrèvement de taxe d'habitation, porté par la majorité présidentielle au total en 2018 les remboursements et dégrèvements constitue un manque à gagner budgétaire à hauteur de 28,5 pourcent des recettes fiscales brute, ce taux a augmenté de 5 points depuis 2013, ce qui traduit une politique fiscale qui repose de façon importante et croissante sur des mécanismes de réduction fiscale, dispositif qui se juxtapose à une mutation considérable du modèle de l'entreprise modèle de l'entreprise qui tend à la financiarisation de l'autre économique. La diminution de la taxe d'habitation ne peut laisser ignorer que d'autres mesures prises auparavant diminue fortement les recettes de l'État et aussi les recettes des collectivités territoriales. Je m'arrête sur les impôts d'État les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État continue de bénéficier à 80 pourcent aux entreprises, la montée en puissance progressive du CIC se traduit ainsi dans le projet de loi de finances par un montant record de 20 milliards d'euros, d'euros, hier, on arrive à la somme rondelette de 27 milliards d'euros, j'observe que l'information relative à la répartition géographique des bénéficiaires du CICE n'est pas accessible. Et cette absence de dispositifs de traçabilité et de contrôle et regrettable et même inquiétant d'un point de vue démocratique, ceci d'autant plus que le CICE n'a pas démontré des effets certains le dernier rapport d'évaluation du comité de suivi du conclut même que le dispositif n'a pas eu d'impact mécanique ni sur les investissements, ni sur la recherche et le développement, ni sur les exportations et ni sur l'emploi, le CIC se pose au moins 2 questions: la première, Madame la Ministre, que fait-on du solde positif des entreprises. La seconde l'utilisons-nous pour répondre aux besoins de développement de notre économie ou pour répondre aux appétits en dividendes des actionnaires, pour le moment, il y a une donnée que l'on connaît avec certitude, c'est que 56 milliards d'euros de cadeaux ont été offerts aux actionnaires l'année dernière, pendant ce temps là, on a pu lire les uns et les autres que des experts avaient là. L'idée géniale de parler de geler le SMIC, impôts locaux, les dégrèvements d'impôts locaux appellent plusieurs observations : tout d'abord, la décision du Conseil constitutionnel relative aux modalités de calcul du dégrèvement coûtera 450 millions d'euros en 2018 à l'État, les contentieux qui seront engagés par les entreprises, ce sera Lyon par un coût de 300 millions d'euros en 2017 et 250 millions d'euros en 2018 tandis que la hausse du coût dégrèvement pour 2018 atteindra 300 millions d'euros supplémentaires, j'en viens au dégrèvement de taxe de la taxe d'habitation, que le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission des finances, on observe que le bénéfice de la mesure sera différent selon la localisation du contribuable bien à revenus équivalents, le montant de l'allégement pourra être très différent, je considère la pour ma part, que la solution retenue par le gouvernement n'est pas satisfaisante, elle crée notamment un risque sur les ressources des communes et groupements, elle ne résout pas la question de la vétusté des valeurs locatives et j'estime pour ma part qu'il est nécessaire de mener la révision des valeurs locatives, il aurait également été préférable d'aller plus loin et temps même progressivement avec expérimentation le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction des revenus n'oublions jamais que les contribuables à la taxe d'habitation n'ont en général pas la possibilité de la déduire de leurs impôts sur le revenu, contrairement aux entreprises qui peuvent déduire la contribution économique territoriale qu'elle s'acquitte de la base de calcul de leurs impôts sur les sociétés ou sur le revenu. L'avis de la commission des finances de doit évidemment dominé mon propos, elle vous propose notre commission des finances d'adopter les crédits de cette mission en les minorant de 3,2 milliards d'euros par cohérence avec les amendements adoptés en première partie, permettez-moi un petit mot personnel avec en déboucher une question, un constat : la question, c'est dans leur ensemble, à qui les dispositifs dont nous parlons sont-ils favorables, c'est que depuis 5 ans, on accentue des mécanismes qui n'ont pas fait leur preuves et qui avantages sans contrepartie aucune la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire leurs actionnaires et pas leurs salariés ils avantagent la minorité qui s'accaparent les richesses de notre pays mais pas l'immense majorité qui les crée voilà aussi et, excusez-moi, mais a-t-il personnel, moi je vous proposerai de ne pas voter ces crédits, merci de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à madame Sophie Primas remplacement de Monsieur Alain Châtillon, rapporteur pour avis des affaires économiques. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues mes propos sont effectivement ceux de notre collègue Châtillon Alain Châtillon et rejoindront ceux de Victorin Lurel qui s'est exprimé tout à l'heure sur les participations de l'État, en effet, il nous paraît indispensable et urgent d'ouvrir avec le gouvernement une discussion visant à redéfinir les modalités du contrôle parlementaire sur les crédits du compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, sans s'interdire le cas échéant de modifier sur ce point, la loi organique relative aux lois de finances je constate en effet que les modalités de ce contrôle ne sont pas satisfaisantes sous leur forme actuelle, chaque année, il est demandé au Parlement de se prononcer sur des crédits dont on sait qu'ils sont très largement hypothétique, de fait, les sommes inscrites en dépenses et en recettes sur ce compte dans la loi de finances initiale sont toujours très éloigné des sommes dans la loi de règlement, l'incertitude concerne également la nature des opérations qui seront réalisés dans l'année, puisqu'on ne connaît évidemment pas à l'avance quels titres vont être achetés ou vendus par l'Agence des participations de l'État, l'embarras du Parlement face à la présentation des crédits du compte d'affectation spéciale est encore plus marquée, cette année,

grâce à des cessions de portefeuilles gérés par l'Agence des participations de l'État, il s'agit d'un projet encore très flou, donc nous ne saisissons pas la logique financière et dont la réalisation risque d'obérer fortement les capacités d'intervention future de l'État dans le capital d'entreprises stratégique,

cela nous paraît assez curieux, on ne demande pas au Parlement d'exercer son contrôle mais comme vous l'avez dit de délivrer un blanc-seing, la commission des affaires économiques, a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat pour le reste, Alain Châtillon souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le dossier de l'aéroport de Toulouse-Madame la Ministre, l'État conserve une participation de 10 pourcent du capital qu'il aura la possibilité de céder à partir du 18 avril 2018,

de la région et du département, l'État devra en tenir compte et préciser s'il vous plaît, ses intentions Alain Châtillon, précise qu'il est totalement défavorable à une cession à si l'Europe et demande que des solutions alternatives : soit trouvées, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des finances, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est avec un esprit constructif que je vais aborder les 3 missions. Les 3 missions engagement financier de l'État investissements d'avenir remboursements et dégrèvements et le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, dont le contenu est pour l'essentiel, la conséquence de la politique menée au cours de ces dernières années, voire des dernières décennies. et ne suscite pas de la part du groupe RDSE de critiques majeures et nous approuvons donc les crédits de ses missions, sauf s'ils étaient effectivement profondément modifié par certains amendements cependant leur examen mérite quelques remarques un certain nombre d'interrogations et d'engagement financier de l'État concerne essentiellement la charge de la dette qui représente la quasi-totalité des crédits, celle-ci peut être considéré comme stabilisé à 41 41,593 milliards d'euros et enregistre même une légère baisse de 0 76 cette stabilisation a bien entendu pour origine des taux d'intérêt excessivement bas. Toutefois, l'encours de la dette continue de progresser, devrait atteintes 96,8 pourcent du PIB en 2018 alors que la zone Euro et en particulier l'Allemagne connaissent une trajectoire inverse puisque c'est une trajectoire à la baisse, le besoin de financement progresse également en raison de cette majoration et de l'arrivée à échéance d'un certain nombre de titres émis lors de la crise financière de 2008 2009, cette situation fait peser sur nos finances publiques, un certain nombre de risques dont le plus alarmant, véritable épée Damoclès est celui d'une possible et sans doute probable remontée des taux d'intérêt dans les années à venir, d'où la nécessité Madame la Ministre, de poursuivre et accentuer les efforts pour engager un réel désendettement, il est vrai que ce mot est curieusement utilisée dans les documents budgétaires en affectant des sommes au désendettement de l'État alors qu'en réalité celui-ci n'existe pas, il serait préférable de parler de contribution au remboursement de la dette ou éventuellement de décélération de l'augmentation de l'endettement, mais certainement pas du désendettement puisque lorsque la dette augmente, c'est une notion qui n'est, qui ne correspond pas à la réalité. Cette présentation, donc, est en effet pour le moins, trompeuse, donc, le terme est a minima, impropre à la mission investissements d'avenir, qui trouve ses origines dans les travaux d'une commission, présidée il y a une décennie par messieurs Alain Juppé et Michel Rocard, illustre la volonté des gouvernements successifs, de soutenir de manière dynamique et sélective, les actions porteuses d'avenir pour notre économie, et en même temps, la difficulté de mettre en oeuvre à pigments les mesures d'incitation, d'accompagnement, sélectionnés dans différents programmes, les 3 programmes d'investissements d'avenir ont été intégrés à un grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros dans le budget 2018 se traduira par l'inscription de 1 virgule 0 8 milliards d'euros de crédits de paiement avec une prévision pour la période 2008 2020, 2 4 milliards d'euros de crédits de paiement ces montants sont relativement modestes et ne paraissent pas à la hauteur de l'ambition affichée de doter notre pays d'une économie performante. Dans cette démarche, on ne peut pas réduire une logique de projet à une stricte logique budgétaire cette réflexion vient compléter une analyse très plus détaillée qui été fournies par notre rapporteur sur ce sujet, la mission remboursements et dégrèvements qui regroupe 115 milliards d'euros de crédit est en forte hausse ne 12 milliards par rapport à 2017, cela est notamment la conséquence de la montée en puissance du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE et de la mise en place du dégrèvement Cellatex habitations je ne reviendrai pas sur le dispositif concernant un texte habitation qui a fait l'objet de nombreux débats et échanges au cours de ces dernières semaines et apparemment qui, en France, encore tout à l'heure lors d'un amendement en ce qui concerne Cissé, même si le comité de suivi a du mal à se prononcer, à mesurer ses effets réels, il renforce incontestablement la capacité de nos entreprises à se développer, mais il faut le considérer comme une condition nécessaire mais pas suffisante pour que les entreprises puissent investir et créer des emplois, lors de sa mise en place, il a été fortement critiquée, voire caricaturer pour des raisons différentes, à droite comme à gauche. Il va laisser la place, en janvier 2019, un dispositif de baisses de charges sociales qui fera passer cette mesure, qui avait un caractère conjoncturel et fragile, un statut structurelle et permanente, donnant ainsi une meilleure visibilité au monde économique. Contrairement à ce que disent certains détracteurs cette mutation ne va pas se traduire par une augmentation du coût du travail, ce serait une bien mauvaise connaissent une méconnaissance totale de la comptabilité de l'analyse des coûts, mais elle va effectivement majoré la base de l'impôt sur les sociétés, conséquence d'autant moins pénalisante pour les entreprises que parallèlement, le taux de l'IS comme le gouvernement s'est engagé devrait être abaissée progressivement de 33 à 25 Le dernier point ne compte d'affectation spéciale participation financière de l'État. C'est le support budgétaire de l'État actionnaire, sa particularité de présenter une programmation conventionnellement à l'équilibre dans le but de préserver la confidentialité sur les opérations de cessions ou d'acquisitions à venir afin d'améliorer la fin si j'ai hérité de la démarche, hein, j'adhère à la proposition du rapporteur spécial inscrire dans le bilan du compte un chiffre correspondant à la moyenne des cessions des 3 derniers exercices, cela constituerait au moins un repère, mais la vraie question qui se pose est de savoir quelle est la ligne directrice je conclus du gouvernement en matière de participation de l'État au capital de certaines langues en grandes entreprises et son implication ou non dans des filières stratégiques, il faut bien reconnaître que des signes contradictoires ont été données au cours des derniers mois dans des dossiers sensibles, ceux de STX et d'Alstom, qui affichage 3 lignes du produit des cessions 10 milliards d'euros annoncés en direction d'un fonds pour l'innovation de rupture et aussi pour l'industrie et même d'un milliard d'euros pour le désendettement, permettez-moi de renouveler mon scepticisme voir mon opposition à ce type d'affichage qui peut être présenté comme une démarche de clarté, mais comme je l'ai évoqué précédemment devient plutôt un facteur de confusion. En conclusion, au-delà de notre approbation de la confiance que j'accordance domaine au gouvernement, je souhaite, Madame la Ministre, vous puissiez dans les mois à venir répondre interrogation que je viens d'exprimer, je vous remercie. de passements est assez significatif. Monsieur Didier Rambaud pour la République en marche pour 6 minutes. Monsieur le Président Madame la la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord, Madame la ministre, si votre pour votre 1ère entrée au Sénat nous a paru peut-être un peu rude, je partage la un peu d'énervement, mes collègues mais je vous adresse néanmoins tous mes voeux de réussite dans vos nouvelles fonctions, nous devons examiner ce matin 3 missions et et 12 programmes, ils ont tous été présentés à avec esprit de synthèse peut-être rapidement, mais avec l'esprit de synthèse et brio par les rapporteurs, qui m'ont précédé, je m'arrêterai tout d'abord au au programme 117 charges de la dette et trésorier de l'État, le niveau d'endettement public, c'est-à-dire le le montant de dette publique rapportée au au produit intérieur brut a augmenté jusqu'à s'approcher du seuil de 100 d'après la programmation pluriannuelle, il est de 96,8 pourcent en 2017 tandis que d'autres pays s'étaient engagés à avoir un ratio de dette inférieure à 60 pourcent du PIB et un difficile inférieure à 3 points de PIB, la France a laissé filer son déficit et sa dette en contradiction avec les règles élémentaires de politique économique contracyclique, se privant de marges de manoeuvre, notamment lors de la crise de 2007, je rappelle qu'avant cette crise, l'endettement public était d'un peu plus de 64 pourcent, c'est-à-dire 64 pourcent en haut de cycle, en réalité, les gouvernements successifs ont fait le choix de laisser se dégrader le niveau d'endettement pour des raisons diverses, mais qui n'échappe pas aux citoyens qui n'échappe pas aux citoyens, notamment quand il observe le sort fait au PLF PLF SS au Sénat et je rappelle le creusement de 7 milliards déficits au citoyen quand il observe la oncle longue liste d'intérêts particuliers que beaucoup ici se sont fait rapporteur toutefois la rapporteur spéciale l'indiquer les crédits alloués à la charge de la dette sont malgré la progression de l'endettement public relativement stable, en légère baisse, pour être précis et s'élève à 41,593 milliards d'euros si la charge de la dette est stable, c'est bien parce que les taux auxquels la France emprunte sont à un niveau historiquement faible, le rapporteur général en en commission des finances a a pointé le risque que ferait courir la hausse des taux sur la soutenabilité de la dette publique, ce risque est néanmoins tempéré déjà parce que la France a profité de la faiblesse des taux d'intérêt pour allonger l'échéance de sa dette, c'est-à-dire que parce que la dette publique présente aujourd'hui une maturité assez longue, une hausse des taux d'intérêt ne devrait pas se traduire immédiatement par une hausse des intérêts à verser, je fais reposer mon propos sur l'étude d'Olivier Blanchard, l'ex-chef économiste au FMI et Zettel meilleur paru en juillet dernier pour le Peterson Institute, il s'appuie sur l'exemple du Japon

à ces conditions et je le cite : une hausse de 200 points de base des taux d'intérêt se traduit par une hausse des paiements d'intérêt de 0,6 pourcent de PIB, la première année et 1 pourcent sur les 2 premières années d'autre part, et vous savez, les taux d'intérêt augmentent, si la croissance et l'inflation augmente dans un telle qu'à l'accroissement du PIB nominal réduira mécaniquement les ratios d'endettement non seulement la politique monétaire de la Banque centrale européenne continue d'être accommodante mais les prévisions de la croissance française nous font écarté l'hypothèse d'un écart entre la croissance française et les taux d'intérêt, quoi qu'il en soit, les pistes évoquées par le rapport spécial sur la mission engagement financier de l'État sont toujours d'actualité, notamment la mutualisation d'une partie de la dette des États membres de la zone Euro pour éviter toute écart entre les taux de croissance et les taux d'intérêt de la Banque centrale s'est par ailleurs au sein de cette mission que le programme 336 porte la dotation en capital du mécanisme européen de stabilité pour un total de 16,3 milliards d'euros répartis en 3 versements ce mécanisme permanent qui a pris la suite du Fonds européen de stabilité financière s'appuie sur le capital apporté par les États membres pour emprunter sur les marchés financiers avec une capacité d'intervention porté à 700 milliards s'il l'a prouvé son utilité comme mécanisme de gestion de crise, il faut désormais sa transformation en off en un fonds monétaire européen, c'est en tout cas le souhait du président de la République qui est en ligne avec les recommandations de Jean-Claude Junker et de la Commission, il s'agirait de sortir de cette logique assurantielle du mécanisme européen de stabilité pour assurer enfin une coordination macro-économique au niveau de la zone Euro, une telle proposition, part d'un constat simple une politique insoutenable dans un État-membre déstabilise l'ensemble de la zone, ce fonds monétaire européen permettrait aussi de clarifier l'architecture actuelle des organes qui interviennent dans la politique économique de la zone Euro, enfin, il s'agirait d'aligner les politiques économiques sur les exigences contemporaines d'économie à la frontière technologique sans transition, c'est aussi l'objectif de la mission investissements d'avenir que nous et qui examinons aujourd'hui dans le cas de la loi de finances initiale pour 2017, elle traduit budgétairement le 3ème programme d'investissements d'avenir et ses 3 priorités : c'est l'objet des programmes de la mission, contrairement à l'an passé, la mission se voit doté de crédits de paiement, il ne s'agit plus d'affichage politique mais d'actions, le programme d'investissement connaît par ailleurs une réorientation, le pays a été ainsi intégrés dans le grand plan d'investissement présenté le 25 septembre dernier l'objectif. Le crurent. Un choc ocre et de doper la croissance du PIB, décline, se décline en priorité pour conclure et je crois que s'il est un point commun : ces 12 programmes que nous examinons, c'est bien cette prise en compte des besoins d'une économie à la frontière, comme la France, merci. Merci, la parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la ligne démission autorisées pour 2018 et de 195 milliards d'euros en dette de moyen et long terme, dont 120 vont d'ailleurs être mobilisés pour amortir la dette existante, je ne parle même pas ici des émissions de bons du Trésor, destiné à assurer les dépenses courantes bons du Trésor dont le taux moyen est d'ailleurs depuis quelques temps, assez proche de 0, comment expliquer cette dette de moyen long terme que je qualifierais de sorte de rentes perpétuelles des marchés financiers sur la France qu'est-ce qui fait le déficit cette année 25 milliards composé de 21 milliards pour le CICE et 6 milliards pour le site la suppression de l'impôt sur la fortune, va coûter 4 milliards de mieux et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique va ajouter 1 virgule 3,4 milliards tout laissant penser, hélas, que la facture sera plus élevée, je pense, notamment, mais, chers collègues, la bagatelle de 30 milliards d'allégements de cotisations patronales qui alourdiront encore cette facture et, même si celles-ci sont engagés pour un tiers environ par la hausse mécanique de l'impôt sur les sociétés, nous avons, en ajoutant les mesures lésinent zozote rien moins que 50 à 55 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales car le problème est là, ce n'est pas pour le développement du Patrimoine collectif de la nation, que l'État s'endette c'est pour conforter et renforcer les patrimoines privés les impôts de tous au profit de quelques-uns, une forme de hold-up d'un nouveau Style, si ces mesures fiscales diverses destinées à la compétitivité des entreprises et de notre économie avait encore un petit peu d'efficacité, cela se saurait, mais je crains que le spectacle accablant des inégalités sociales grandissantes dans notre pays de la précarisation du travail du sous-emploi chronique des bas salaires, constitue une démonstration éclairante de l'échec des politiques suivies jusqu'alors la dette en soi, cela n'a rien de répréhensible, car qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'économie sans crédit, rappelons que si la dette publique pèse aujourd'hui environ 100 pourcent du PIB, la dette privée et celle des entreprises et des ménages se situent entre 140 et 150 pourcent et qu'elle pose autant de questions, tout doit être fait dans notre pays pour que l'appréhension de la finance sur l'activité économique soit au plus limitée qu'il s'agisse de l'État comme des entreprises et de nos concitoyens l'intermédiation financière oui mais sans épuiser ou capter toute la valeur ajoutée, ceci posé, quand un pays s'endette pour réaliser telle ou telle infrastructure porteuse d'avenir, ce peut-être une ligne ferroviaire à grande vitesse ou un canal fluvial essentiel à la transition écologique et à l'amélioration des flux de transport de marchandises dans notre pays, il choisit une dette porteuse de future source de progrès et de développement quand ils s'endettent pour payer la suppression de l'impôt sur la fortune, l'allégement de la fiscalité du capital et surtout amortir des décisions budgétaires antérieurs, nous ne sommes plus dans une logique vertueuse qui peut nous dire à quoi serviront demain les 4 milliards perdus de recettes d'ISF, il est temps de mettre en oeuvre un grand effort de réflexion citoyenne dans notre pays, celui d'un audit citoyen de la dette en toute transparence pour séparer le bon grain de l'ivraie et nous libérer de la soumission à la loi des marchés financiers, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Claude Malhuret pour les indépendants pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues Il est paradoxal et un peu triste que nous examinions conjointement les crédits de la mission engagement financier de l'État et investissements d'avenir, le montant de crédits dédiés à la première révèle, en effet, le poids du passé qui obère nos politiques publiques aujourd'hui et pèsera demain sur les épaules de nos enfants, la seconde est un effort salutaire mais modeste en comparaison pour préparer l'avenir de notre économie et de notre société, le programme 117 de la mission engagement financier de l'État, qui représente la quasi-totalité des crédits de la mission contient la charge d'intérêts de notre dette souveraine dans un contexte de taux très faibles, cela a déjà été rappelé ces crédits sont en légère baisse, ils atteindront tout de même 41,6 milliards d'euros en 2018, soit le 2ème poste budgétaire de l'État, c'est 6 fois le budget de la justice, ou encore 10 milliards d'euros de plus que le budget de la défense. Cette diminution conjoncturelle de la charge de la dette ne doit pas masquer ce fait inquiétant, la dette française continue de s'accroître inexorablement alimentées par des déficits qui ne se résorbe que trop lentement. Les efforts consentis par le gouvernement vont dans le bon sens mais il nous paraissait insuffisant pour combler notre retard sur les autres pays de la zone Euro et en particulier sur l'Allemagne, notre trajectoire de désendettement, par exemple, est nettement en deçà de celle de nos voisins, en 2016, la dette publique française représentée 96,3 pourcent du produit soit un écart de 28 points de PIB en 2022, selon les estimations de la commission des finances du Sénat. L'écart sera de 39 points de PIB avec l'Allemagne, approchant les 50 pourcent d'endettement, ce différentiel sera sans précédent dans l'histoire récente de l'Europe, il ne doit pas être sous-estimé, il augure une perte d'influence durable de la France face à des partenaires ayant des marges de manoeuvre plus importante et par conséquent pour agir et pour décider. Si nous ne parvenons pas à maîtriser plus sérieusement les dépenses de l'État qui ont progressé de 20 pourcent entre 2007 et 2016 si nous ne parvenons pas à résorber nos déficits effectif et structurelle de façon plus volontaire si enfin et, en conséquence, nous ne parvenons pas à diminuer notre stock de dettes de manière forte, c'est bien notre stature politique en Europe et dans le monde qui en pâtira, il ne s'agit pas ici que de chiffres, mais bien de la capacité du politique à agir encore au service des Français et des valeurs de la République. Pour conclure sur cette dimension, Madame la Ministre, nous pouvons vous reprochez le niveau actuel d'endettement de l'État qui n'est pas de votre fait, mais bien une télé française qui dure depuis 30 ans, nous pouvons seulement vous conseille d'adopter une démarche plus volontaire alors qu'une fenêtre d'opportunité exister risque peut-être de se réformer prochainement, profitant de la conjoncture favorable pour assainir en profondeur nos finances publiques et relancer notre économie, nos voisins européens le font, vous le faites plus timidement, nous souhaitons vous aider à le faire plus fort. Parce qu'il en va de l'avenir de notre société et notre économie, il en va de la qualité de vie que nous les grands à nos enfants à ce sujet, les crédits de la mission investissements d'avenir nous rendent plus optimistes, il regroupe des programmes du même nom que nous devons à l'Intelligence de 2 hommes, Alain Juppé et Michel Rocard qui ont oeuvré ensemble dans leur rapport, pour préparer la France aux défis de demain. Les programmes d'investissements d'avenir ont précisément pour objet d'augmenter la croissance potentielle de la France en misant sur l'économie de l'Intelligence, l'innovation et la recherche, ils seront intégrés au grand plan d'investissement voulue par le président de la République leur montée en gamme tant quantitatif que qualitatif doit être salué, mais il gagnerait à être mieux articuler avec les initiatives européennes en la matière, comme par exemple le plan Junker. Dans un grand nombre de domaines, la masse critique requise d'investissement viendra en effet d'une Europe plus solidaire et plus volontaire à l'architecture renouvelée, c'est ce que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France appelle l'Union de financement et d'investissement qu'il nous reste à bâtir ensemble. Le groupe, les indépendants votera les crédits de ses missions pour saluer l'orientation défendue tout en espérant Madame la ministre, avoir encore plus de raisons de les voter l'année prochaine, je vous remercie. Merci, cher collègue Monsieur Michel Canivet pour le groupe Union centriste en remplacement de Nathalie Goulet pour 6 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, malgré l'heure tardive à laquelle nous sommes arrivés, il s'agit de l'examen 2 missions qui sont particulièrement importantes d'une part en terme de volume financier qu'elle représente et aussi parce qu'elle traite à la fois du passé de la gestion de de nos finances publiques et elle prépare aussi l'avenir, c'est donc essentiel que nous puissions nous attarder un peu sur les différentes missions qui sont proposés en tout cas, le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à ce que nous ayons une gestion la plus rigoureuse possible de nos finances publiques, la traduction que l'on trouve dans la manière de dont TGV gérer nos finances publiques ces dernières années, c'est l'état de la dette, tout le monde la connaît parfaitement, nous sommes à plus de 2200 milliards de tonnes d'près de 1800 à la charge directe de l'État, nous sommes proches des 100 pourcent du PIB donc il importe que nous puissions agir très rapidement pour que cette dette puisse se réduire, en tout cas il faudra Madame le ministre, que nous puissions en 2000 dès 2018 et dans les Budgets à venir s'attacher à réduire le déficit public puisque c'est la seule façon de pouvoir effectivement réduit à l'état de la dette, or on le sait bien, le déficit public pour 2018 sera supérieur à celui qui est prévu en 2017 de façon significative, quand même, puisqu'il avait été prévu à 70 milliards en Lot financier initial et sera 76 et devrait être à 83 l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire, on le sait bien, les recettes supplémentaires qui peuvent être générés par une croissance qui repart ne seront pas suffisantes pour pouvoir atténuer ce déficit, il importe donc que nous puissions aussi réaliser un effort sur la dépense publique qui est, je le rappelle, la plus élevée au parmi les plus élevés de l'Union européenne, c'est dire que le chemin que nous avons à faire en la matière et quelques pistes ont déjà été esquissée dans le budget 2018 sur le logement, les contrats aidés, enfin la mission travail notamment, mais cela ne ne suffira pas et parmi nos sujets d'inquiétude, il y a bien entendu celle de la dette, les intérêts de la dette, je vous le rappelle, représente un peu plus de 40 milliards l'année prochaine, paradoxalement, quand on regarde l'évolution des intérêts de la dette ces dernières années, depuis 2014, les intérêts de la dette pour diminuer malgré l'augmentation du de la quantité d', c'est-à-dire que nous avons pu profiter de taux d'intérêts extrêmement bas, mais chacun le sait bien, ici, c'est que la situation risque de ne pas durer et il importe donc que nous puissions agir en la matière et je vous rappelle aussi que, en 2018, la France sera après l'Italie, le plus gros emprunteur de l'Union européenne sur les marchés, il faut aussi que nous puissions être assurés de pouvoir trouver les moyens de financement de l'ensemble de notre dette, si l'on veut que notre note financière ne soit pas dégradée, c'est dire le chemin qu'il reste à parcourir là dessus alors un autre volet de de ce que nous examinions ce soir porte sur la question de l'État actionnaire, effectivement, c'est extrêmement important, on sait bien que l'application de l'État a permis de maintenir dans notre pays a un certain nombre de fleurons 7 dernières années, nous ne sommes pas au niveau du groupe de l'Union centriste pour une intervention forcenée de de l'État dans l'économie, mais parfois, il importe que nous puissions y recourir il faut que l'on sache aussi à cet égard, pouvoir se séparer de nos participations, le moment venu, parce que l'État n'a pas n'a pas de nature à devoir maintenir des participations, donc nous souhaitons à cet égard, Madame la Ministre, savoir quelle est véritablement la stratégie de l'État en la matière est-ce que c'est effectivement d'essayer de se procurer des revenus supplémentaires par les dividendes qui sont octroyés ou est-ce que c'est simplement une participation des participations stratégiques pour pouvoir maintenir des fleurons économiques dans notre pays, autre point sur la question de l'État actionnaire qui taraude le le groupe de l'Union centriste sur la question de la cohérence de l'intervention publique en matière d'actionnariat, aujourd'hui, l'actionnariat vers vers le les entreprises est partagée entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence des participations de l'État, pour nous, il est extrêmement important que celle-ci soit effectué de façon cohérente, c'est-à-dire qu'il y a une vraie vraie stratégie, une unité qui défini, donc il importe que l'on puisse travailler pour que l'on soit assuré que l'ensemble de ces outils à la disposition de l'État est une démarche qui soit parfaitement cohérent, donc la la définition de de la stratégie

concernant les investissements et le soutien aux investissements dans notre pays, il importe néanmoins Madame la ministre, que l'on puisse trouver la traduction dans les projets de budget qui ne se présenter ici, nous avons à déplorer que les crédits de paiement soit extrêmement limitée au regard des engagements du pays à 3, ça veut dire qu'il y aura sur les exercices à venir des efforts extrêmement importants à mener, or on sait qu'en terme de recherche, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, puisque nous sommes loin de l'objectif défini par la stratégie de Lisbonne en 2000 et nous avons donc un un vrai effort à faire là dessus, enfin sur la question des dégrèvements qui est aussi une question importante, je voudrais rappeler l'attachement du groupe de l'Union centriste à la notion de crédit impôt recherche, nous considérons qu'effectivement dans notre pays, c'est un outil absolument essentiel, dire que on encourager et entreprises, donc merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci monsieur Martial Bourquin pour le groupe socialiste, pour 7 minutes. minutes. Ce président, madame la ministre, chers collègues, ce compte d'affectation spéciale participation financière de l'État s'illustre par l'incertitude et la confidentialité qu'ils en tout. Et cette incertitude cette confidentialité conduisent à progressivement dessaisir le Parlement de son pouvoir de contrôle sur la stratégie de l'État, le chiffre annoncé de 5 milliards inscrits en recettes, comme ce fut le cas ces dernières années sur le compte, participation financière de l'État et plus qu'hypothétique, cependant nous pouvons constater un infléchissement qui nous paraît extrêmement préoccupant. Cet infléchissement est perceptible sous 2 aspects à la fois dans les déclarations du ministre de l'économie, mais surtout dans ses dernières décisions ainsi Bruno Le Maire déclaré au mois de juillet, je cite, à partir du mois de septembre, nous allons céder des participations non stratégiques de l'État dans un certain nombre d'entreprises publiques, encore faut-il, madame la ministre d'avoir la même définition du terme stratégique et permettent un véritable débat démocratique au sein du Parlement, en effet, le recentrage du portefeuille de l'État a des participations de l'État implique que le gouvernement précise sa conception de l'État stratège et cette redéfinition du périmètre de l'État actionnaire ne saurait intervenir sans un véritable débat au Parlement. Sinon. Le pouvoir de contrôle du Parlement est complètement mise sous tutelle sécession, selon le ministre devrait atteindre 10 milliards d'euros pour permettre le financement de l'innovation. Et plus précisément l'innovation de rupture, alors permettez-moi, même la ami de souligner ici un 1er aspect de cette stratégie, il reviendrait en effet à céder 10 pourcent du portefeuille de l'État pour abonder un dispositif qui représenterait 2 pourcent des montants consacrés chaque année à l'innovation, de même, ce serait ignorer que ces cessions consiste pour l'État français à se priver de dividendes qui entre 2012 et 2016 Selver à 3,26 milliards d'euros versés au budget général à titre de comparaison, les crédits proposés par le projet de loi de finances 2018 pour la mission, relations avec les collectivités territoriales et de 3,66 milliards d'euros. Dans les récentes décisions du ministre qui ont consisté à céder le 5 septembre dernier 4,5 pourcent du capital d'énergie, puis le 2 novembre dernier 4 73 pourcent du capital de Renault sécession présentée comme les premières étapes du plan de cession d'actifs alors une 1ère question peut se poser, si 1,5 milliard provient de ses 2 récentes sessions, il reste à savoir où trouver l'et 8,4 milliards pour alimenter ce fonds de l'innovation, ce sont donc des entreprises publiques qui risque était directement visé, nous voudrions en savoir plus, ici, avant de voter ce chapitre important du budget de la nation, outre ce fonds de l'innovation, un des autres objectifs poursuivis par le comté le désendettement de l'État le rapporteur monsieur Châtillon disait que ça représente une charge annuelle de 2,5 Et que les participations ont une rentabilité courante de 3,5 pourcent ça reviendrait à une absurdité financière on perdrait de l'argent l'État avec ses stratégies perdrait de l'argent alors que cette décision pourrait pareil d'une logique financière extrêmement douteuse, elle correspond surtout à une menace et c'est ça d'essentiel sur la capacité de réaction de l'État face aux difficultés sectorielles en la soumettant aux contingences budgétaires annuelles à rebours d'une vision à l'enterrement l'industrie ça ne peut pas être que du court terme, ça doit être du Moyen et du cours du et du long terme, je souhaite revenir par exemple sur un épisode en 2012 PSA enregistrer une perte historique de 5 milliards d'euros. Son action en bourse, passer de 80 euros à 5 euros. L'État agit dans le capital de PSA avec Dongfeng et aujourd'hui cette société redresser. Qu'est-ce qu'a fait Barack Obama lorsque l'automobile américain General Motors était en difficulté. Ils ont nationalisé en partie. L'automobile américaine et-il redresser. Et c'est là que notre interrogation, comprenez est entière, c'est que, quelle place pour l'État stratège aujourd'hui dans la politique du gouvernement sur la fusion Alstom-Siemens le refus du gouvernement d'entrer au capital empêche le gouvernement de jouer un rôle stratège le prive d'exercer tout contrôle Direct sur ce nouveau groupe qui va se constituer, il aurait mieux valu certainement que Siemens et moins de 51 pourcent et que l'État français et un droit de regard et puisse agir sur cette fusion pour faire un EADS du ferroviaire, voilà nos interrogations, je pense que compte le ministe Bruno Le Maire, était interrogé sur ces questions, il nous a dit que la politique de l'État, c'était avant tout des baisses de charges et il nous a très peu parlé de cette vision de l'État stratège qui, de la Libération Charles-de-Gaulle jusqu'à maintenant une vision où l'État français. Entend jouer un rôle dans l'économie pour faire en sorte que lorsqu'une entreprise est en difficulté, ou lorsqu'il y a une volonté de faire en sorte qu'un secteur industriel soit dopé, hé bien l'État puisse jouer tout son rôle, j'ai l'impression que dans cette vision purement financière à court terme, hé bien ça risque de se traduire par une conception de l'État stratège rabougri. Merci, cher collègue, la parole est à madame Delphine Gény-Stéphann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances pour 10 minutes.

monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je commencerai tout d'abord par vous assurer de mon plein respect de vos débats de nos discussions dans cet hémicycle, je crois que c'est important. J'aurais bien aimé moi aussi que, en effet, nous soyons dans des conditions un peu meilleure pour discuter et une heure différente mais ça n'est pas de de mon fait, et soyez assuré de mon plein respect pour ce débats je vais commenter successivement les différentes missions programmes et et comptes spéciaux qui sont à l'ordre du jour. Ce soir tout d'abord la mission engagement financier de l'État qui fait l'objet d'un rapport spécial de madame le sénateur Nathalie Goulet, au nom de votre commission des finances, qui recouvre les crédits nécessaires à l'État pour assurer son financement en toutes circonstances l'essentiel des crédits de la mission concerne le programme 117 la charge de la dette et de la trésorerie de l'État pour 41,2 milliards d'euros. Avec Madame, le rapporteur spécial, plusieurs d'entre vous se sont exprimés sur l'évolution de la dette publique et je vous remercie de votre appel à la ville, vigilance collective quant au niveau de la dette et à l'évolution des taux d'intérêt, la période de taux d'intérêt très bas, voire négatifs dont notre pays bénéficient depuis plusieurs années sous l'effet d'une politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne ne durera pas éternellement, la BCE s'est engagé au cours des derniers mois dans un resserrement monétaire progressif, même si le rythme de ce resserrement restera tributaire de l'affermissement de la croissance en Europe et du retour graduel de l'inflation dans ce contexte, notre estimation de la charge des intérêts de la dette intègre de façon prudente et raisonnables cette remontée des taux à moyen terme, conformément aux orientations fixées par le président de la République, ce projet de loi de finances pour 2018 constitue une première étape dans l'affermissement de la crédibilité budgétaire budgétaire et financière de la France, ce renforcement de notre crédibilité passe en 1er lieu par la mise en oeuvre des réformes structurelles indispensables à notre économie et permettant une modernisation de nos services publics, il passe en second lieu, par la réduction du poids de la dépense publique et la baisse des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et les ménages. à cet égard la progression, la progression ininterrompue de la dette publique depuis la crise de 2008 connaîtra un coup d'arrêt l'an prochain avant une inversion de tendance nette prévue sur l'ensemble du quinquennat sur 5 ans, la dette publique serait ainsi ramené à 91,4 pourcent du PIB en 2020, 2 contre 96,8 pourcent prévu pour la fin de l'exercice 2017.

le président de la République a affirmé que cette mutualisation correspondant à des engagements pris séparément par les tous les États-membres n'est pas politiquement acceptable ni pour la France ni, ni pour la pour les autres États-membres. Par ailleurs, s'agissant du traitement prudentiel des titres souverains, nous sommes opposés à toute évolution, renforçant les exigences en capital associé aux détentions de dette souveraine. S'agissant de notre position vis-à-vis des agences de notation, je veux sur ce point vous rassurer au second semestre 2017, les 3 principales agences de notation, Standard dames poursuite et Moodys ont confirmé la notation soient double asseoir à de de la France, ces notations témoigne de la qualité de la signature française et, depuis l'Automne 2016 ces notations sont associés à une perspective stable. Je passe maintenant au 4 autres programmes de la mission peut F. tout d'abord le programme 114 les appels en garantie de l'État, vous avez évoqué Madame la rapporteurs le sujet des engagements hors bilan, j'observe que le travail mené depuis la levée de 2006 en matière de recensement des engagements hors bilan a significativement contribué à la sincérité des comptes de l'État aujourd'hui, la France dispose en matière d'engagements hors bilan d'une information riche et fiable. Pour autant, les enjeux et montants mis en valeur par la comptabilité générale incite à adopter une logique de surveillance active, ainsi que le recours systématique aux règles de l'actuariat. Grâce à la gestion active de ses engagements, les crédits du programme 114 sont en réduction continue. Pour 2018, ils augmentent sous l'effet de l'inscription de 63 millions d'euros au-dessus des procédures de soutien financier au commerce extérieur, qui n'avait pas fait l'objet d'actes d'inscriptions de crédits en 2017 dans le cadre d'un tour du transfert à BP assurance export de la mission précédemment assuré par la Coface, cette réforme qui fait de la BPI là-dessus, l'interlocuteur public privilégié des entreprises pour leur financement va dans le sens d'une meilleure efficacité d'un moindre coût, tant pour les entreprises que pour les finances publiques. Le programme 145 épargne retrace les primes d'épargne logement versée par l'État lors de la mobilisation de comptes d'épargne logement ou de la clôture des plans d'épargne logement le gouvernement parachève cette année, la réforme de ce dispositif. lot pour RAM 168 majoration des rentes retrace les crédits destinés au remboursement partiel des majorations droite légal et de de rente bien j'ai pourcent 41,8 millions d'euros. presque 65 ans de remboursement des majorations de rente par l'État au débit rentiers, les objectifs de politique publique ayant justifié initialement dépenses ont atteint, il est proposé de mettre un terme au dispositif proposition de bonne gestion, qui a reçu le soutien de votre commission des finances qui a elle proposé un amendement permettant d'améliorer le dispositif. Enfin, le programme 344 fonds de soutien relatifs aux prêts contrats financiers structurés à risque et destiné au financement du fonds de soutien en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant souscrit des emprunts structurés et instruments financiers sensibles, le gouvernement n'est pas favorable, madame la pape rapporteur spécial à la réouverture de ce guichet. S'agissant des comptes spéciaux je passe rapidement sur le compte spécial, participation de la France au désendettement de la Grèce, l'engagement de ces crédits se fera dans un cadre européen en fonction de l'issue du 3ème programme grec qui court jusqu'à l'été 2018, le comte de concours financiers avance à divers services de l'État, organisme gérant des services publics enregistre il est convenu d'appeler France du Trésor pour l'essentiel, il s'agit du préfinancement des aides communautaires de la PAC, qui sont, et donc ces actions sont neutres dans le déficit. J'en viens maintenant au compte d'affectation spéciale participation financière de l'État qui a fait l'objet de beaucoup de de remarques ce soir et d'un rapport spécial du ministre Victorin Lurel au nom de votre commission des finances, et dans le rapport pour avis du sénateur du sénateur Alain Châtillon, je les remercie, ainsi que l'ensemble des intervenants, des intervenants Depuis 2015, l'État actionnaire a fortement fait respirer son portefeuille en menant une politique particulièrement dynamique de cessions et d'investissement. Cette politique était était orientée vers la protection des intérêts essentiels de notre économie, il s'agit par exemple de la restructuration des secteurs stratégiques avec les recapitalisations récentes d'EDF ou Areva, il s'agit de peser dans les négociations permettant de préserver le savoir-faire et l'emploi en France. Avec le cas STX et il s'agit aussi d'avoir une action stratégique dans le domaine ferroviaire avec un rapprochement européen de 1er plan entre Alstom et Siemens. S'agissant de l'aéroport de Toulouse qui a été évoqué, je voulais préciser qu'aucune décision n'est prise à ce jour concernant l'exercice par l'état de son option de vente, l'État prendra sa décision au cours des prochains mois, en recherchant le meilleur intérêt de l'ensemble des parties prenantes à ce dossier.

au défi des transitions économiques industrielle, technologique et écologique, il est sans doute nécessaire d'être plus sélectif en matière d'actionnariat public. Le gouvernement souhaite donc désormais conduire le recentrage de ce portefeuille sur 3 axes prioritaires. Le premier, les entreprises stratégiques qui contribue à la souveraineté de notre pays, en particulier dans le domaine de la défense et une du nucléaire 2ème axe les entreprises participant à des missions de service public ou d'intérêt je générale camp l'électorat ne détient pas de levier non actionnariat suffisante pour préserver les intérêts publics et le 3ème acte le 3ème axe, ce sont des interventions dans des entreprises lorsqu'il y a un risque systémique, une respiration du portefeuille de l'Agence des participations de l'État est ainsi envisagés afin de répondre aux mutations qui viennent bousculer le monde économique et notre tissu industriel, nous aurons l'occasion de préciser ses grandes orientations en temps utile et la représentation nationale sera bien entendu associée à cette réflexion. Vous avez mentionné nécessaire d'actifs et la dotation d'un fonds pour l'innovation, à hauteur de 10 milliards d'euros, conformément à l'engagement du président de la République, ce fonds préparera l'avenir de notre économie en n'investissant sur des novation ou l'État, et même en partenariat avec des investisseurs privés d'assumer une partie des risques technologiques de long terme qu'il convient de prendre pour réussir, nous travaillons mécanismes et aux dispositifs qui permettront d'un point de vue technique et juridique d'enfer n'objet utile. Ce fonds doit être opérationnel début 2018 et pour commencer, il sera alimenté en numéraire par une part du produit des récentes cessions des participations dans J. Renault le solde sera constitué de participations publiques n'ayant pas vocation à être cédé, mais versant des dividendes réguliers ces participations seront sortis du fond au fur et à mesure que l'abondement numéraire tirés des cessions montera en puissance. Le rendement annuel de ce fonds de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros par an sera sanctuarisée, pour garantir notre effort annuel en matière d'innovation, en effet, il nous faut notamment pour des innovations dite de rupture, retrouvez le temps long nécessaires. Pour flécher ses ressources vers les projets les plus prometteurs,

d'investissement dans l'innovation dans l'économie de la compétence et dans la transition écologique, il est également question avec la mission investissements d'avenir qui a fait l'objet d'un rapport spécial de votre commission des finances. Rappelons que le 3ème programme d'investissements d'avenir, a été lancée avec l'ouverture de 10 milliards d'euros d'autorisations d'engagement 2017 le PLF 2018 prévoit l'ouverture des premiers crédits de paiement avec un peu plus d'un milliard d'euros de crédits de paiement. Maintenant ministre, il serait bon de de conclure parce que il y a, il y a encore un certain nombre d'amendements qui sont à examiner.

Pour terminer, j'aborderai la mission remboursements et dégrèvements qui fait l'objet d'un rapport spécial, l'enveloppe de crédit global de ces 2 programmes est très importante puisqu'elle est d'environ 100 milliards d'euros pour le 1er le programme 200 et 15 milliards pour le programme de

Voilà, donc j'ai entendu aussi parler de la réforme de la taxe d'habitation, mais je pense que j'ai traité l'essentiel des sujets qui avaient été abordés ce soir, et donc je vous épargne la fin de ce discours. Si Madame la ministre, voilà donc nous en avons fini pour les interventions donc. Sur le crédit, la mission engagement financier de l'État, il n'y a pas d'amendement dont je vous demande de le vote genèse au cette mission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. L'article 55 pardon. Oui, Monsieur le président de la commission des finances. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, maintenant que la demi-heure d'interruption de milieu de soirée va peser un peu lourd puisque nous devrons arrêter impérativement à une heure 30, reprenant demain avec d'autres programmes à 10 heures et demie du matin, donc nous avons 9 heures d'interruption obligatoire, donc il reste une dizaine de minutes pour une dizaine d'articles et cet je pense que c'est un peu Mission : Impossible, voilà la difficulté qui explique sans doute l'état d'esprit de mes collègues ce soir donc je le regrette, il faudra que nous reprogrammer Lyon j'irai sans doute vendredi irai la fin l'examen de de ces de ces crédits mais j'invite évidemment mes collègues à une très grande j'irai concision dans l'expression, si l'on veut essayer néanmoins d'avancer le plus possible.

C'est article vise à supprimer Madame Nice, mes chers collègues, un engagement pris par l'État depuis 1949 qui consistait à majorer légalement les rentes AGR de retraite, c'est finalement un engagement qui avait pour objectif notamment après guerre, de protéger les assurés bénéficiaires de ces contrats de la forte inflation qui existait à l'époque, l'État rembourse ainsi chaque année une partie des majorations légales de rente viagère versée au cours de l'année précédente par les assureurs et rembourse aux personnes physiques ayant souscrit ou adhérer à une assurance, et ça pour les rentes viagères avant 1980 cette ce mécanisme de revalorisation consiste concrètement à demander aux assureurs de préfinancer les majorations légales auprès des assurés, l'État remboursant ensuite aux assureurs c'est ce remboursement de l'État aux assureurs que propose de supprimer l'article 50 5, or l'exposé des motifs du projet de loi de finances 2018 précise qu'il s'agit d'une aide financière apportée écoutez bien aux assureurs pour tenir leurs engagements contractuels, or ce n'est pas aux assureurs mais aux assurés. Que c'est d'être financière s'adresse, je l'ai dit, à l'heure au nom de la solidarité nationale, il convient de noter que ce système de majoration de rente viagère a été instituée en dehors de toute clause contractuelle et de réglementation du code des assurances, l'article 55 transfert ainsi intégralement une charge publique aux assureurs, destiné pourtant à l'origine au financement de mesures de solidarité découlant de l'intérêt général, je précise enfin que la Cour des comptes, dans la lettre adressée au ministre de l'économie, le 21 juillet dernier estime jusqu'à l'extinction du contrat à 1,8 milliard d'euros, le montant du transfert sur un nombre réduit d'entreprises d'assurance, le déficit des finances publiques, justifie certes de faire des efforts, mais justifient difficilement l'élaboration de ce type de mesures immédiates et confiscatoire qui présente d'ailleurs un risque d'inconstitutionnalité. Oui, Monsieur le Président, la commission vous propose un retrait au profit de l'amendement suivant qui lui propose, non pas le de de se désengager de sa mais de prévoir un étalement des provisions sur 6 ans. Merci madame la ministre. Oui, comme indiqué à l'instant donc, le gouvernement souhaite la suppression du du dispositif de participations de l'État au financement des majorations de rente viagère et donc est défavorable aux premières amendement revanche favorable à l'amendement proposé par le rapporteur général. Merci madame la ministre Monsieur sont il est retiré. le je vais le retirer, je note simplement que, comme souvent, on fait confiance à la parole orales prononcées par le ou la ministre de l'occurrence par vous, Madame la Ministre, j'espère en tous les cas que cette parole sera tenu puisque c'était une relation de confiance, je note enfin que lors de l'examen à l'Assemblée, cette mesure n'avait semblé poser aucun problème, mais ça l'avait même pas été examinée sexe avait été rejetée, je note donc dans la navette parlementaire cette utile de rappeler parfois un certain nombre de fondamentaux, donc à l'égard des assurés et des assureurs, je vous remercie de la proposition que vous faites, notamment au travers de l'amendement, qui est présenté par le rapporteur général et donc je retire mon amendement. Merci Monsieur sont donc le 636 rectifier, donc qui est un étalement sur 6 ans de ces dispositions qui est défendue donc par la commission des finances, qui a reçu un avis favorable de de la ministre de Madame la ministre du gouvernement qui est pour, pas l'même Cohen pour explication de vote excusez-moi. pas je vais pas expliquer le le le vote mais je veux quand même protesté solennellement par les les conditions de travail d'examen là parce que je trouve ça inadmissible on est épuisé, finalement, là vous nous demandez d'aller à toute vitesse de rajouter un quart d'heure, c'est pas des conditions, on est très peu dans l'hémicycle et franchement ce n'est pas digne des législateurs que nous sommes. Merci Madame Cohen donc. Sur sur le 636 rectifier, donc qui est l'amendement de la commission qui a eu reçu un avis favorable du gouvernement, qui est un étalement sur 6 ans, on peut passer au vote. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. L'article 55, ainsi amendé. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous poursuivons avec l'article 55 bis, un amendement 300 de Madame Goulet, au nom de la commission des finances présenté par monsieur monsieur le président, ma dans la ministre oui c'est un amendement qui concerne un rapport qui a été demandé au gouvernement sur les PEL et donc sur les sur l'épargne logement et et il est proposé d'élargir le le le l'amendement non pas à l'examen de la prime d'État, mais à l'ensemble du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement.

Qui est corrompu. Qui s'abstient, il est adopté, donc article 55 bis même vote. Donc il est adopté. Après l'article 55 bis, l'amendement 137 rectifier bis madame de Romilly. Oui, merci Monsieur le Président, conformément aux statistiques publiées par l'INSEE, le marché de l'ameublement et dépendant de celui de l'immobilier depuis 3 ans, il a ainsi chuté de 10 pourcent provoquant de nombreux sinistres économiques et sociaux tenta fabrication quand distribution spécialisée d'ameublement en l'absence de toute perspective de reprise de l'activité immobilière, les 125000 salariés de la filière meuble françaises sont menacés et nécessitent pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d'incitation à la consommation de meubles ainsi cet amendement propose afin de soutenir la consommation française d'ameublement et les emplois induits d'autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l'achat de meubles, cette mesure de déblocage temporaire en partielle et partiale de l'épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles et donc à la croissance avec les enfants, les rentrées fiscales induites dans la TVA, le secteur de l'ameublement domestique est exclusivement concernés par cette mesure pour mémoire des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 96 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Merci, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, la Commission a proposé un retrait de cet amendement, considèrent qu'il complexifie rétro, le dispositif du PL, alors que nous souhaitons le rendre plus lisible. Merci madame la ministre. Merci Michel, président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, cette proposition n'apparaît pas opportune, le plan d'épargne logement est un produit destiné à favoriser une épargne régulière par les ménages, leur permettant de constituer un apport personnel et d'obtenir un prêt à taux fixe, fixé à l'avance, pardon, dans le cadre d'un projet immobilier, le fonctionnement du produit ne permet pas d'effectuer un retrait sur leur plan afin d'acquérir des meubles me en à usage non professionnel untel retrait au cours de la vie du plan serait contraire à la logique même du produit, c'est pourquoi nous proposons de retrait sinon moi j'ai.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, le Fonds monétaire international, en complément de son activité principale d'appui aux États en situation de crise de balance des paiements, appuie les pays à faible revenu par des prêts aux concessionnaires cette activité qui s'est fortement développé à la suite de la crise de 2008 2009 et réalisée pour l'essentiel à travers à travers la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, la contribution française à cet effort prend aujourd'hui la forme de prêts de la Banque de France à la fr PC garanti par l'État, le dernier prêt accordé date de 2010 pour 1,3 milliard de droits de tirage spéciaux, soit environ 1,5 milliard d'euros, le FMI a sollicité ses États-membres pour renouveler et amplifier leur contribution, la France soutient pleinement cet effort renforce et en matière de promotion du développement et de lutte contre la pauvreté dans ce cadre, il est prévu que la Banque de France accorde un nouveau prêt d'un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux, soit environ 2,4 milliards d'euros au taux change actuel le présent acte article vise à autoriser l'État a apporté sa garantie à ce prêt.

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Je mais au bois le les crédits compte spécial, participation de la France au désendettement de la Grèce. Qui est pour. Qui est quand. Qui s'abstient, il était et sont adoptés. Je mais au les crédits du compte spécial participation financière de l'État qui est pour.

Oui, le c'est le prix, là je voudrais juste dire que je vais voter contre cet article 68 en effet, il demande que le il y a un rapport au Parlement sur les autoroutière avec la rentabilité la distribution faite aux actionnaires, or, en 2014 et 2015 en tout Jean-Jacques Filleul et moi-même nous avons travaillé sur le rapport à la suite de du rapport de de du duperie dans la serre de l'autorité de la concurrence sur le problème des autoroutes et décidé de confier à l'Arafer le soin de contrôler les autoroutes, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un article de loi qu'en se demandant des rapports au Parlement il y a qu'à demander à l'Arafer de faire son travail de, de, de, de présenter les rapports concernant la rentabilité des autoroutes et les destructions des des actionnaires et, par conséquent, je voterai contre l'article 68. Merci, cher collègue Madame Cohen pour explication de vote. Tout à fait, Monsieur le Président, à l'opposé, nous avons voté en faveur de cet article 68 car il pose une question tout à fait pertinente, celle du devenir des entreprises jadis public ici la part détenue par l'État dans les sociétés d'économie mixte de concessions autoroutières qui ont été privatisées, le fait, le fait est que la privatisation des autoroutes a constitué lorsque l'opération s'est produite une des décisions publiques les plus critiquables les plus critiqués des 15 dernières années, et les choses ne se sont d'ailleurs pas arrangé, notamment pour les usagers victimes de la hausse des péages cette article 68 et donc parfaitement bienvenue et devrait nous inspirer pour d'autres, sur la situation, par exemple, les Liens plus ou moins ténue entre politiques, industriels et maîtrise publique qui se sont assez largement évanouie dans les opérations de privatisation pour examiner autre exemple intéressant, quels ont été les conséquences réelles de la privatisation par tranche de l'opérateur historique de téléphonie, à savoir Orange et de la libéralisation des télécommunications sur la qualité de service rendu et l'appareil économique du pays, en général, tardive ou très matinale et donc nous voterons cet article. Merci. On peut passer au vote non Monsieur Lurel postulation de vote très courte. Chers collègues. Il avait émis un avis me semble favorable puisque ce texte issu, il me semble, l'Assemblée nationale, ça n'a pas été remis en cause en commission des finances était un avis favorable. La commission des finances n'a pas donné d'avis sur l'article 68 mais il n'a pas donné non plus d'avis défavorables. Alors donc jamais au bout article 68 qui est pour. Levez bien la non. Est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 68 là que l'amendement 416 qui le défend.

on essaye de passer très vite et c'est dommage, malgré tout, cet amendement est un amendement d'appel à partir de 2012, l'État s'est dotée d'une doctrine de l'état actuel actionnaire cette doctrine a été progressivement confortée avec par exemple l'instauration du droit de vote double ou une nouvelle gouvernance des entreprises à participation publique, or cette doctrine de l'État actionnaire qui avait l'Avantage de donner une ligne claire à l'intervention de l'État dans les entreprises qui semble aujourd'hui être remise en cause. En 1er lieu en renonçant à exercer l'option d'achat des titres à hauteur de 20 pourcent du capital d'Alstom, lors du récent rapprochement entre Alstom et Siemens, le gouvernement a mis en pratique une nouvelle conception du rôle de l'État actionnaire, beaucoup plus restrictive que la précédente, il se prive ainsi de la possibilité d'orienter sur le moyen ou le long terme, les choix stratégiques de cette entreprise qui concerne aussi la préservation de l'emploi, en second lieu, en décidant de céder 10 milliards de titres pour alimenter un fonds de financement d'innovation, le gouvernement diminue drastiquement les actifs de l'État au bénéfice de qui aura lieu cette cession massive de titres, je vous pose la question : un ancien ministre interrogé également sur la pertinence de s'engouffrer dans la brèche déprimé désertion qui n'aurait d'autre effet que d'appauvrir l'État actionnaire, je cite : quand j'entends dire que la situation des finances publiques conduirait l'État à céder les participations, je crains que ce ne soit là un prétexte pour céder à quelques amis des parts de société, fin de citation, c'est ce même c'est ce même ancien ministre qui faisait remarquer que vendre des participations de l'État ne créait pas de recettes budgétaires, et on le sait, au vu de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt, les rendements du placement de ces 10 milliards seraient bien plus faible que les dividendes qu'il rapporte aujourd'hui à l'État, Il est tard, on aimerait y voir plus clair, Madame la Ministre, et surtout comprendre la nouvelle doctrine s'il y en a une, de l'État actionnaire, le ministre de l'Économie a en effet déclaré et on a auditionné ici dans le cadre de la commission économique que le rôle qu'on a fait jouer à l'État jusqu'à présent n'était pas le bon, d'accord, mais le Parlement doit être, doit en être informé et ce compte d'affectation spéciale pour nous, nous en dire plus sur les choix opérés et à venir sur la réelle stratégique de l'État actionnaire. Dans le rapport pour avis le rapporteur fait homme. Alors il faut conclure, chers collègues, là il faut conclure là je veux dire, 2 minutes 30 et sont écoulées, je suis désolé, à cette heure-ci, on peut pas de dépasser. Oui, alors je je comprends qu'ils sont d'accord, on a quand même accepté une demi-heure. Merci, merci, merci, je remercie, je donne la parole non terminé, je donne la parole pour l'avis de la commission c'est Monsieur Lurel rapporteur spécial. Qui est un avis favorable, Madame la Ministre. Pour le gouvernement. Merci monsieur le président Clinton, Monsieur le Sénateur, donc je comprends que certains un amendement d'appel qui a donc appelle une discussion qu'un peu plus large, d'une part sur donc les les conditions dans lesquelles s'effectuent les les sessions à la perte de majorité par l'État au capital d'une entreprise publique, je rappelle que le cadre légal et réglementaire prévoit déjà que, pour la plupart des grandes entreprises, en fait, le, le Parlement doit autoriser cette cette privatisation est qu'il est pas parfaitement impliqué dans la décision généraliser une pratique de consultation de la représentation nationale, comme cela est proposé par un rapport préalable sur les privatisations des de tout type d'entreprise détenue majoritairement par l'État, Marc n'apparaît pas opportun, par ailleurs, monsieur le sénateur, vous avez souhaité une clarification sur la stratégie d'intervention de l'État en tant qu'actionnaire dans les entreprises, je crois que enfin le le gouvernement est vraiment assez Net dans ses choix, il s'agit de rester actionnaire des entreprises stratégiques qui contribue à la souveraineté de notre pays dans les entreprises qui participent à des missions de service public ou d'intérêt général, quand l'État ne peut pas par des leviers non actionnariat préserver les intérêts publics et ensuite avoir la capacité d'intervenir dans des entreprises lorsqu'il y a un risque systémique et donc nous préconisons le retrait de cet amendement. Merci Monsieur Hurel, rapporteur pour la commission. Je je vous entends, nous rappelons que si je devais avoir 10 milliards même si le 1er ministre vient de changer, devant le Conseil national de l'industrie, il faudrait céder un tiers des participations dites ses cibles. 100 des participations globale et totale de l'État sur 100 milliards de l'APE 10 milliards c'est 10 pourcent et sur le périmètre véritablement cibles dans le secteur concurrentiel, ça représenterait un tiers, on ne pourra pas céder en l'espace d'une année, 10 milliards réduit aujourd'hui après sa déclaration à 8 milliards qui seraient des prêts de titres fait je ne sais que à quelle instance paix ne peut, on ne peut pas recevoir de dividendes ces dividendes seraient versés, je ne sais quel fonds sur quelle ligne vous quel programme il y a là un mystère qu'il faut clarifier, c'est la raison pour laquelle il y a 3 entreprises qui font l'objet d'une loi, là c'est une loi parce qu'on ne peut pas descendre en deçà de 70 pourcent pour certains ou de 50 pourcent pour d'autres, ces 3 entreprises, pour le reste, il faudrait lorsque l'État fait une opération qui consiste à lui faire perdent la majorité au sein des conseils ou ramener Fluence, ce qui a déjà des titres à votre double d'informer le Parlement d'informer le Parlement de toute façon, la presse, le souverain, il y aura pas la de délit d'initié, il y aura pas de d'information donnée au marché qui pourrait, si j'ose dire, déstabilisé les cours et donc brader le Patrimoine de l'État, il me semble qu'il faut trouver un compromis raisonnable entre la confidentialité qui doivent entourer ces opérations et la nécessaire information du Parlement et de l'autorisation que nous délivrons et ça, ça paraissait en compromis, c'est un un amendement borné.

on a, on a prouvé, en gros, on va dire à la lettre l'article 68, là nous sommes en total désaccord avec l'esprit, la lettre de cet article 69, il nous sommes c'est un article qui manque de vision à long terme qui ne peut manquer d'inquiéter. Pour aller très vite, nous pensons qu'il s'agit de faire de l'Agence des participations de l'État, une sorte de club d'investissement dont la seule fonction serait de réaliser des cessions de titres et de réclamer un retour sur investissement sur les titres détenus en clair, madame la ministre, il nous semble que la paix deviendrait une sorte de boursicoteurs public dont la qualité serait mesurée à la hauteur des plus-values et là peut-être qu'il y a un petit problème, ça rejoint d'autres éléments qui sont d'une lice pulsions, évidemment, on s'occupera pas des stratégies à l'oeuvre derrière on va ramasser la la plus-values tirées des cessions et des dividendes remontée des entreprises détenues donc devenu opérateurs de l'État, la paix aussi même peut-être un contrat d'objectifs et de moyens tendant assurer entre session rémunération du capital au niveau de des recettes non fiscales au budget de l'État résumer, vous avez un portefeuille de 100 milliards d'euros en valeur boursière ou non de types divers, vous devez nous rapporter cette année 4 milliards ou bien 5, si ça marche encore mieux, peut-être 6 cette vision de la propriété, qui par réaction de sociétés, nonobstant leur nom ou leur valeur absolue ou relative n'est pas la nôtre, il nous semble que l'APE ne doit pas seulement être un demandeur de titre opportuniste ou pour présenter un peu quand même Astor là de du dormant.

Il est adopté. Genèse au voix les crédits du compte spécial accords monétaires internationaux qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. Je mets au bois, les crédits compte spécial avant diverses, services de l'État organismes gérant du service public qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. Je mais on voit les crédits de la mission Investissements d'avenir. Et pour qui est contre.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, l'objet de ces thèmes cette. Amendement et de tirer les conséquences de 2 amendements adoptés lors de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2018, il convient de minorer les crédits du programme 201 remboursements et dégrèvements d'impôts locaux de 3 milliards 206 millions d'euros en autorisation d'engagement comme en crédits de paiement, en effet, l'amendement 97 a supprimé, article 3 sur le dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce qui minore les remboursements et dégrèvements du programme de 40 millions d'euros, l'amendement 99 à supprimer, quant à lui, l'article 3 ter qui prévoyait un dégrèvement pour certains contribuables ce qui minore les remboursements et dégrèvements du programme 201 266 millions d'euros, par ailleurs, compte tenu des décaissements otite du contentieux sur la taxe de 3 pourcent sur les dividendes, il convient de majorer les crédits du programme 200 remboursements et dégrèvements d'impôts d'État 700 millions d'euros, soit la différence entre les 5 milliards d'euros décaissements prévus et les 300 millions d'euros initialement provisionné dans le projet de loi de finances pour 2018.

Donc c'est un amendement de constatation, tout le monde connaît bien les 2 sujets là qui justifie cet amendement de de constatations puisque c'est lié à une décision de la majorité sénatoriale qui a été suivi d'un vote majoritaire, donc voilà, donc c'est un amendement de constatation, bon ça étonnera personne, on a des heures de débat derrière nous et chacun a et chacune à respecter la légitimité les arguments des uns et des autres, donc au nom de la commission des finances, je donne un avis favorable a-t-il personnel,

quand entre. Qui s'abstient. Il est adopté et donc jamais au bois le les crédits de la mission remboursements et dégrèvements qui est pour. Qui est contre. Ils sont adoptés. Chers collègues, je vous remercie d'être resté jusqu'à 7 heure très tardive ou très matinale en fonction lors du jour du jeudi 17 décembre la séance reprendra 10 heures 50 à 14 heures 30 et le soir : suite du projet de loi de finances pour 2018 examen démission Agriculture Alimentation forêt affaires rurales économie outre- mer, recherche et enseignement supérieur, la séance est levée.